La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du vendredi 27 septembre 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. en application de l'article 28 de la Constitution, la session ordinaire de 2019-2020 est ouverte. M. Charles Revet a fait connaître à la présidence qu'il se démettait de son mandat de sénateur de la Seine-Maritime à compter du 30 septembre 2019, à minuit. En application de l'article L.O. 320 du code électoral, il est remplacé par M. Pascal Martin, dont le mandat de sénateur a commencé aujourd'hui, à zéro heure. En votre nom à tous, je souhaite la plus cordiale bienvenue à notre nouveau

avons terminé avec le débat sur la régression de la place de l'agriculture française sur les marchés internationaux et les conséquences en termes de qualité et de protection du consommateur de produits importés qui ne correspondent pas aux normes françaises. Mes chers collègues, nous allons Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je vous rappelle que l'auteur de la demande du débat dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, qui aurait pu penser que la force exportatrice de la France puisse un jour être remise en question ? cette question, nous pouvons désormais nous la poser. Avec un excédent de la balance commerciale agricole divisé par deux au cours des cinq dernières années, on peut aujourd'hui affirmer que, si nous n'y prenons pas garde, nous constaterons notre premier déficit en 2023

puisse devenir totalement dépendante des importations de l'agriculture d'autres pays ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes et témoignent malheureusement d'un déclin de notre agriculture, déclin que nous sommes les seuls à connaître au niveau mondial. En effet,

Elle est passée de la troisième place en 2005 à la sixième place aujourd'hui. Lamentable ! Quant à l'Allemagne, elle a progressé, alors que l'Espagne et les Pays-Bas se maintiennent. Au même moment, de nouvelles puissances émergent, telles que la Pologne, le Brésil, la Chine et l'Inde. Les raisons de ce déclin sont multiples. Je n'en citerai que trois, qui démontrent tous les « défauts » de notre pays. pays. Les trois quarts de cette érosion s'expliquent par un effet de compétitivité négatif dû, premièrement, au dumping social des pays européens concurrents- le coût horaire du travail est, en France, 1,7 fois plus élevé qu'en Espagne et 1,5 fois plus élevé qu'en Allemagne ; conséquence : le kilo de porc coûte 10 centimes de moins en Allemagne qu'en France, par exemple. les charges de production connaissent une augmentation plus élevée en France, de 4 % à 7 % entre 2016 et 2019. L'alimentation animale, les engrais, l'énergie, les produits phytosanitaires coûtent plus cher qu'ailleurs, et la loi pour l'équilibre des relations une tendance à la surréglementation accentuée. Nous surtransposons sans cesse les normes européennes- dernier exemple : le glyphosate, autorisé cinq ans en Europe, sera interdit

classe ainsi la France comme le pays où le degré d'exigence est bien supérieur aux autres en matière de normes environnementales. Et comme si cela ne suffisait pas, nous en rajoutons une couche tous les jours : les zones de non-traitement ne sont, en la matière, que Tous ces éléments, jumelés à l'agri-bashing, conduisent sans relâche à la perte de notre capacité de production. En laissant penser aux Français que notre agriculture n'est pas vertueuse, nous dégoûtons de plus en plus les producteurs, créant ce mal-être insupportable pour les agriculteurs. Quelle profession accepterait de travailler dans cette ambiance délétère, qui conduit un agriculteur à se suicider tous les deux jours ? Eh oui ! Tout cela entraîne un recours massif à l'importation de produits agricoles que nous pourrions très bien produire chez nous ! Bien sûr ! Depuis 2000, les importations ont ainsi presque doublé. Les chiffres sont désespérants : un fruit et un légume sur deux sont importés ; l'importation de produits laitiers a été multipliée par deux entre 2005 et 2017 ; l'importation de volaille a connu une hausse de 37 % sur la seule année 2017

Ces importations portent sur des produits bas de gamme et nous les retrouvons surtout en restauration hors foyer. Elles représentent 60 % à 80 % de la viande de volaille et 75 % de la viande bovine. À ce propos, je souhaite faire une parenthèse sur un concept à la mode que vous défendez, monsieur le ministre : la montée en gamme. Si nous n'y prenons pas garde, cette montée en gamme se traduira par la coexistence de deux sortes de consommateurs

sur la qualité sanitaire des produits importés : les éléments du rapport du groupe d'études sénatorial démontrent qu'un quart des produits importés ne respecte pas nos normes, chiffre édifiant qui atteste de « notre » naïveté ! Autre risque : celui de scandales alimentaires. Comment expliquer au consommateur que la France doit changer de modèle et que ce changement passe par la consommation croissante de denrées importées du bout du monde pour la production desquelles on a utilisé des produits interdits chez nous ? Le risque de voir s'accélérer la hausse des volumes importés existe également : en effet, tous ces éléments favorisent un écart de compétitivité qui fera que les produits importés seront moins coûteux que ceux qui sont produits en France,

enfin de ne plus connaître l'autosuffisance alimentaire, alors que nous savons que la planète comptera bientôt 9 milliards d'habitants, ce qui fait craindre d'éventuelles pénuries alimentaires. Il faut sauvegarder notre autosuffisance alimentaire et refuser d'entraîner, par démagogie verte, Pour conclure, je voudrais, monsieur le ministre, vous rappeler la phrase célèbre d'un de vos prédécesseurs, le surintendant Sully, prononcée en 1604- nous ne nous ne retenons souvent que le début de cette citation, mais la suite est dans la droite ligne du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui : « Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée, les vraies mines et trésors du Pérou ». perspective, Sully proclame la liberté du commerce des grains et abolit un grand nombre de péages. Il ouvre de grandes voies de communication et fait creuser plusieurs canaux, dont le canal de Briare, qui relie la Seine à la Loire. Il pousse les paysans à produire plus que nécessaire

Les décisions de demain sur les normes, sur les traités de libre-échange, seront lourdes de sens et auront des conséquences irréversibles sur l'avenir de la France. Il est vraiment temps de conclure,

tous ensemble, pour qu'elle n'atteigne pas la France. Au bout du compte, le cours du porc, qui était à 1,10 ou 1,15 euro, est monté à 1,60 euro et pourrait atteindre 1,80 euro ; nous exportons en Chine, et c'est très bien ! Mais il faudrait faire pareil pour la viande

Dans les restaurants, en France, il y a en gros 75 % à 80 % de viande étrangère ; dans la restauration hors domicile, ce chiffre est encore plus important. Si, en nous bagarrant, comme nous souhaitons le faire, nous arrivons à changer cela,

pour que l'agriculture française ne se retrouve pas en grande difficulté par rapport à nos concurrents. Troisièmement, je pense qu'il faut éviter d'opposer compétitivité, d'une part, exigence environnementale et sociale et qualité, d'autre part. Cette opposition me paraît passéiste.

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

collègues, le 14 mars dernier, la Cour des comptes européenne a une nouvelle fois pointé du doigt les faiblesses des systèmes de contrôle et de surveillance des produits bio, révélant que seuls 40 % de l'ensemble des produits bio analysés au niveau de l'Union européenne et provenant de pays tiers ont pu voir

de la consommation et de la répression des fraudes constatait que 17 % des contrôles physiques sur les produits issus de l'agriculture biologique importés de pays tiers étaient « non conformes » en 2017.

J'aurai deux questions. Premièrement, alors que la stratégie française semble consister en un alourdissement toujours plus important du cahier des charges des produits agricoles français, comment comptez-vous garantir que chaque denrée alimentaire destinée à la consommation humaine ou animale en provenance d'un pays tiers corresponde strictement aux standards français et européens de production ?

À quelles conditions le haut niveau d'exigences normatives demandé aux agriculteurs et aux industriels de l'agroalimentaire français peut-il contribuer au développement de nos exportations ? C'est la question générale qui vous est posée, monsieur le ministre, et je voudrais l'illustrer à partir de certains enjeux du CETA. Pour les producteurs et les industriels, la prise en compte des normes sanitaires et environnementales des produits échangés est fondamentale dans le modèle alimentaire européen. Elle est un facteur important de la compétitivité française. Par exemple, s'agissant de la sécurité sanitaire et phytosanitaire et du respect du principe de précaution, les bovins, au Canada, sont nourris de fourrages composés notamment d'ingrédients interdits dans les élevages européens : des hormones, des farines animales, des antibiotiques activateurs de croissance et des OGM.

européenne a rappelé que le niveau de protection de la santé de sa population ne pouvait être compromis, et que le principe de précaution devait être respecté, la tentation est forte de ménager les partenaires commerciaux, d'édulcorer ou de reporter des mesures ambitieuses pour la sécurité et la santé des consommateurs européens. Afin de préserver et de développer les positions à l'export de l'agriculture et de l'agroalimentaire français, comment et sur quels points, monsieur le ministre, le Gouvernement entend-il faire des concessions sans sacrifier les principes de qualité et de protection auxquels sont attachés nos concitoyens ?

car il s'agit d'un dispositif normatif qui touche à la qualité des produits agricoles et alimentaires. J'attire également votre attention sur le risque que pourrait constituer la nouvelle gouvernance de la PAC en matière de subsidiarité

monsieur le ministre, mes chers collègues, cela a été dit, l'agriculture française souffre d'une concurrence que l'on peut qualifier de déloyale de la part de pays moins exigeants sur le plan tant social qu'environnemental. Une part bien trop importante de notre alimentation est importée, avec des conséquences sur la qualité des produits et sur les revenus de nos agriculteurs. Pour autant, la réponse ne peut en aucun cas résider dans l'affaiblissement de notre réglementation qui protège à la fois la qualité de notre alimentation, notre environnement, mais aussi la santé tant des citoyens que de nos agriculteurs. Au contraire, je fais partie de ceux qui défendent le renforcement de ces exigences. Selon moi, une part de la solution à la problématique posée aujourd'hui réside dans la relocalisation de l'alimentation. Il s'agit d'une attente sociétale profonde, qui a besoin d'être soutenue et accompagnée par les pouvoirs publics. Or on constate trop souvent des signaux allant dans le sens contraire. Le vote du CETA par l'Assemblée nationale en fait partie : les accords de libre-échange entraînent, on le sait, une course aux prix toujours plus bas et au moins-disant. À l'opposé, les projets alimentaires territoriaux constituent, j'en suis convaincu, un outil efficace pour créer des dynamiques de relocalisation. Ces projets alimentaires territoriaux sont encore trop peu nombreux et souffrent d'un manque de moyens. Pourtant cette animation territoriale est plus que jamais nécessaire, notamment depuis que la loi Égalim prévu un objectif de 50 % de produits de qualité et de 20 % de bio en restauration collective d'ici à 2022. Monsieur le ministre, ma question est la suivante dans le cadre du prochain projet de loi de finances, soutiendrez-vous une augmentation significative du budget des projets alimentaires territoriaux, notamment en vue d'atteindre les objectifs de la loi Égalim concernant la restauration collective ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nos concitoyens sont aujourd'hui de plus en plus attentifs à leur mode de consommation. Ils souhaitent pouvoir contrôler et maîtriser les produits dans leur assiette, en connaissant leur provenance et leur mode de production. L'étiquetage des produits a été une avancée considérable. Il a permis d'assurer une traçabilité effective selon des normes françaises et européennes. Il a également permis de sécuriser le consommateur dans ses choix. Depuis quelque temps, les applications mobiles fleurissent parallèlement pour répondre à ce besoin d'information et de traçabilité. De consommateur à « consomm'acteur », la responsabilité sociale et environnementale de notre consommation est devenue un acte citoyen. Grâce à des outils divers et variés, le consommateur s'émancipe des produits et des modes de vie que le marché avait pu concevoir pour lui. Il devient autonome dans ses choix et contribue à la régulation de la société de consommation. Il devient un véritable acteur de marché. Ma question, monsieur le ministre, est la suivante : comment pouvons-nous accompagner nos agriculteurs et nos producteurs face à cette révolution numérique tout en respectant le choix du consommateur d'être informé ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, s'il y a bien un secteur où la France n'a pas à rougir d'être comparée à ses voisins, c'est bien l'agriculture. Notre pays est de loin le premier producteur de l'Union européenne pour la production tant végétale qu'animale. Nous devançons largement l'Allemagne et l'Italie, nos deux principaux compétiteurs européens. L'image de l'agriculture française et de notre agroalimentaire est excellente à l'étranger. Elle contribue au rayonnement international de notre pays. Notre filière dégage depuis plusieurs décennies des excédents qui soutiennent notre balance commerciale, laquelle demeure malheureusement structurellement déficitaire. Comme l'aéronautique, la chimie et le luxe, la filière agricole donne à la France de solides arguments à faire valoir sur la scène internationale. Cependant, cette position se fragilise et la situation se dégrade dangereusement. Alors que nous étions encore troisième exportateur mondial il y a quinze ans, nous avons rétrogradé à la sixième place. Ce recul s'articule en outre avec une augmentation continue et significative des importations, notamment intra-européennes. À ce rythme, la France pourrait connaître son premier déficit commercial agricole en 2023. C'est parfaitement impensable ! Il est urgent d'enrayer cette tendance avant que notre agriculture ne décroche pour de bon. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour améliorer la compétitivité de notre agriculture, et pour lutter contre les surtranspositions de normes européennes et les mesures franco-françaises qui freinent notre compétitivité ? À quand un choc de compétitivité pour soulager nos agriculteurs et leur permettre de lutter à armes égales avec leurs homologues européens ? Nos agriculteurs n'ont pas peur de la compétition, mais ils veulent pouvoir concourir avec les mêmes règles ou à tout le moins avec des règles équitables

dégrader. Le Président de la République nous a donc demandé de travailler à la mise en place du pacte productif, notamment pour les industries et les entreprises agroalimentaires, qui ont d'énormes problèmes à la fois en termes de recrutement et pour avancer. Menonville, notre volonté n'est pas de peser sur les agriculteurs. Nous voulons que la compétitivité soit la plus forte possible. Nous travaillons à l'échelle européenne afin que l'Europe monte en gamme dans la même direction que nous. Nous avons fait un pas sur les travailleurs détachés il y a un an et demi,

Férat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que la France était le second exportateur mondial de produits agricoles dans les années 1990, elle se place aujourd'hui à la sixième place. Les parts de marché détenues dans le monde sont passées de 7,7 % en 2000 à 4,8 % en 2015. Ainsi, la France affiche en dix ans le plus fort recul mondial ! Or certains concurrents européens directs de la France maintiennent leur position, tels que l'Allemagne et les Pays-Bas. Je n'évoquerai pas le CETA ou le Mercosur. Je ne rappellerai pas les surtranspositions des normes en France ni les surcroîts de charges et de contraintes administratives subies uniquement par les Français. Je veux rappeler avec force le rôle primordial des consommateurs pour soutenir les agriculteurs, les éleveurs et les viticulteurs français. Même si la désinformation va grandissant entre l'agri-bashing et les approximations scientifiques des journalistes en herbe, les consommateurs doivent savoir que la France a la meilleure agriculture du monde ! L'indice de durabilité alimentaire a donné en 2018 à la France la note de 76,1 sur 100,

J'ai par exemple signé la pétition européenne « Eat original » afin de rendre obligatoire la mention d'origine sur les produits alimentaires. Enfin, j'estime que laisser à des produits étrangers, qui ne respectent pas les normes environnementales ou sociales imposées à nos agriculteurs, le libre accès à nos étals est une concurrence déloyale. Si on joue au même jeu, mais pas avec les mêmes cartes, la partie est perdue. Seulement, il ne s'agit pas de jeu, car tous les deux jours un paysan français se suicide

! Ma question est simple : que comptez-vous faire pour que ces distorsions de concurrence, inadmissibles à l'intérieur même de l'Europe, cessent de s'accentuer, non seulement parce que certains pays prennent du retard, mais aussi parce que nous voulons bouillir plus blanc que blanc !

des difficultés rencontrées par les hommes et les femmes qui ont choisi de travailler dans ce domaine. Confrontés aux normes européennes, aux contraintes environnementales, aux coûts de la main-d'oeuvre et du matériel, à la concurrence déloyale des filières informelles et à l'absence de contrôle de la qualité des produits concernés, aux difficultés de trésorerie, à la lourdeur et au caractère contraignant de la réalité administrative, aux risques naturels majeurs, aux maladies répétées et successives de nombreuses filières- bovine, volaille, porcine ... -qui ont contribué à l'élimination intégrale de cheptels, aux problèmes sanitaires qui en ont

de tout détruire. En effet, vous avez décidé d'éliminer l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, l'Odéadom, malgré les difficultés et le recul de notre agriculture. Monsieur le ministre, quelles sont vos ambitions pour l'agriculture française en général, et celle des outre-mer en particulier ? La parole

En termes de prix, nous serons toujours plus chers que les autres pays du fait de charges trop lourdes, du coût de la main-d'oeuvre, du prix des mises aux normes et des carburants, etc. etc. Pourtant, s'il y a bien un domaine dans lequel l'agriculture française est compétitive, c'est la qualité de ses produits ! Les normes françaises, il est vrai souvent contraignantes et surtransposées, assurent la sécurité alimentaire et le respect des êtres vivants. Elles garantissent aussi une agriculture utilisant moins de produits phytosanitaires qu'ailleurs. Il est donc plus que nécessaire de communiquer sur la qualité de nos produits et d'afficher distinctement la provenance des aliments. Cela nécessite de clarifier l'étiquetage, lequel doit être lequel doit être lisible et transparent pour les consommateurs, en particulier sur les produits transformés. Il est vendeur d'afficher la provenance française des aliments ; même les industriels

Pour qu'un produit soit estampillé « Fabriqué en Aveyron », il faut qu'au moins 50 % des matières premières proviennent de ce département. Ainsi, les consommateurs qui achètent des produits sous ce logo sont certains de la provenance de leurs achats. par cette action d'achat, ils soutiennent l'emploi des agriculteurs, des producteurs et des transformateurs du département. Vous comprenez, monsieur le ministre, que l'étiquetage des produits peut tout changer pour notre agriculture. Envisagez-vous de de faire évoluer les pratiques sur l'étiquetage des produits et surtout des produits transformés ? La parole est à M. le ministre.

et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Égalim, précise un certain nombre d'interdictions en matière de consommation humaine ou animale. Or la production française est loin de satisfaire nos besoins alimentaires, à l'instar d'ailleurs de la production européenne. Alors Alors que chaque Français consomme en moyenne 9 kilos de pâtes par an, nous importons massivement du blé dur, faute de semences adaptées et de surfaces agricoles dédiées. Ce blé dur est acheté par les industriels de l'agroalimentaire prioritairement au Canada, premier producteur de blé dur mondial. Or vous n'êtes pas sans savoir que le blé dur est pulvérisé à l'herbicide avant récolte, de façon à être plus rapidement récolté. Cette pratique, peu répandue chez nous, est très courante outre-Atlantique. Il en est de même pour les produits d'importation d'origine animale, dont le nombre explose : on enregistre une progression de plus de 87 % en France depuis 2000. depuis 2000. Je vous serais donc reconnaissante, monsieur le ministre, de bien vouloir m'indiquer quel dispositif aux frontières intra et extra-européennes a été mis en place pour garantir aux consommateurs qu'aucun résidu de produits chimiques et de substances interdites n'est présent dans ces produits alimentaires d'importation. mes chers collègues, monsieur le ministre,

il s'érode et notre position au regard des marchés mondiaux se dégrade inexorablement. En 2012, nous occupions la cinquième place mondiale. Sept ans plus tard, nous sommes rétrogradés à la sixième, confirmant par là une tendance de fond qui a débuté, il est vrai, voilà deux décennies et même un peu plus. Cette situation préoccupante a dans un passé récent interpellé le Sénat et conduit à un rapport publié en 2013. Ce n'est donc pas si loin ! Il était apparu alors que l'appareil commercial français aux exportations agricoles et agroalimentaires n'avait pas su s'adapter à l'évolution des marchés mondiaux, à la différence de celui de pays européens qui avaient su bâtir une stratégie et se doter d'outils efficaces d'accompagnement. Voici quelques insuffisances alors pointées du doigt du côté de l'État, une compétence dispersée entre cinq ministères- pour mémoire, un seul ministère est concerné au Pays-Bas ; des opérateurs français qui s'ignorent quand d'autres pays européens agissent en synergie lors des grands salons mondiaux une frilosité des organismes assurantiels nationaux à garantir les PME exportatrices et, très souvent, une absence de conseils adaptés pour celles-ci ; enfin, des inadaptations administratives pouvant constituer des freins et parfois des blocages. Les choses ont-elles changé depuis lors ? Qu'en est-il, monsieur le ministre, de votre analyse de la situation actuelle ? Il faudrait d'ailleurs, d'une manière générale, que les parlementaires soient informés des suites de leurs propositions, à défaut de quoi l'exercice auquel ils se livrent serait d'un intérêt très très relatif et même sans intérêt du tout. Établir une stratégie victorieuse consiste à définir des objectifs et à faire en sorte que les moyens mis en action convergent afin de les atteindre, et pas l'inverse. Quels sont les projets du Gouvernement à l'égard du soutien aux exportations agricoles et agroalimentaires ? En quoi pourraient consister vos initiatives ?

ou au ministère, car nous pouvons les aider dans le cadre d'une stratégie nationale.

Si notre pays maintient sa place de premier producteur agricole dans l'Union européenne, avec une prédominance dans les marchés des céréales et bien évidemment celui du vin, il ne cesse néanmoins de perdre des parts de marché sur le commerce alimentaire mondial, que ce soit pour l'élevage ou les céréales.

troisième rang. Comment avons-nous pu laisser notre agriculture emprunter cette pente descendante ? Les raisons, nous les connaissons en partie : une surabondance de normes réglementaires et administratives européennes et franco-françaises, et un trop-plein de charges qui pèse sur la compétitivité. Je pense surtout que, depuis 2011, les gouvernements successifs ont tout simplement lâché l'agriculture. Aujourd'hui, nos agriculteurs demandent non pas l'aumône, mais des prix rémunérateurs. Or nous sommes dans un système de prix mondialisés avec des contraintes nationalisées et européanisées, qui ne permet ni de tirer profit de la qualité et de la traçabilité de nos produits ni, surtout, de répondre à leur attente en termes de prix.

le bas. S'y ajoutent évidemment les difficultés liées à l'embargo de la France vis-à-vis de la Russie. Pour cela, il faut que la France exige la mise en place en Europe d'un marché boursier destiné aux productions de qualité correspondant à nos normes, pour un marché mondial de qualité. Monsieur le ministre, pouvez-vous être porteur d'un tel projet ? À défaut, quelles sont vos propositions pour permettre à notre agriculture de reconquérir sa place sur les marchés internationaux ?

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la multiplication des accords de libre-échange touchant les produits agricoles inquiète tous nos concitoyens. Les termes de ces accords semblent conduire notre agriculture dans une situation inextricable, où l'on répliquerait hors des frontières de l'Union européenne un principe de libre circulation, sans les garde-fous que la construction européenne vise précisément à garantir. Nous tremblons l'idée d'ouvrir notre table à des pays qui, sur tous les points sensibles pour la compétitivité de nos producteurs et pour la qualité de l'alimentation de nos concitoyens, promettent trop systématiquement de considérables risques, sans les outils de maîtrise que nous nous efforçons avec tant de difficultés de construire en Europe. Jusqu'alors, monsieur le ministre, vous répliquiez que l'on ne peut pas souhaiter exporter en refusant d'importer. C'est un peu caricatural. Pour notre part, nous refusons un cadre où nous devrions importer beaucoup plus pour exporter seulement un peu plus, et voir ainsi s'accentuer le déclin de notre excédent commercial. Nous refusons également des accords qui ne seraient pas assortis de garanties effectives quant aux engagements sanitaires et phytosanitaires qu'ils comportent. Je me bornerai à vous faire deux demandes. La première porte sur la réalisation par l'Union européenne d'un audit sérieux sur les contrôles sanitaires aux frontières réalisés par les États membres, en lieu et place de l'habituelle collection de « fiches pays

Quels sont les gages de sérieux de ce contrôle ? Ma seconde demande est que, face à la considérable dégradation de la position de la France sur le marché mondial des produits agricoles, le Gouvernement s'attache à mettre en place le plus rapidement possible une stratégie complète de reconquête de nos positions. Le Premier ministre a indiqué vous avoir demandé de mandater FranceAgriMer à l'effet d'établir un diagnostic fin sur ce point. Pouvez-vous nous indiquer selon quelles modalités vous entendez associer

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat d'aujourd'hui sur la régression de la place de notre agriculture part d'un constat alarmant. Je tiens à mon tour à féliciter notre collègue Laurent Duplomb pour son rapport d'information sur ce sujet, qui nous permet de nous exprimer afin de défendre nos agriculteurs dans leur travail au quotidien. plus particulièrement aux producteurs de fruits et légumes, qui sont touchés par une concurrence déloyale. Ce thème a déjà été abordé, mais je voudrais parler de deux cas précis : la cerise du Gard et la carotte de Créances, exemples d'une aberration économique, sanitaire et écologique. Certains produits phytosanitaires utilisés sur les fruits et légumes sont désormais interdits en France. Même s'ils sont parfois interdits en Europe, ils peuvent néanmoins bénéficier de nombreuses dérogations. de la cerise. En 2018, les producteurs se sont mobilisés pour dénoncer cet abus dont ils étaient les victimes. En effet, ils n'étaient plus autorisés à utiliser le diméthoate contre la mouche, alors que leurs concurrents étrangers, notamment turcs, pouvaient importer leurs fruits en France. Or, même si la production française n'est pas suffisante, les importations doivent être réglementées pour assurer une concurrence saine.

Aucune dérogation n'était possible, car il s'agissait d'une décision de l'Union européenne, et donc entérinée dans le droit français. Pourtant, certains pays européens, notamment l'Espagne et l'Italie, ont obtenu, semble-t-il, des dérogations. Cette production française est donc frappée de plein fouet par la concurrence déloyale, ce qui a révolté nos agriculteurs. Ils réclament, très légitimement, une réglementation unique pour un marché unique. De plus, il est choquant que l'on accepte de mettre dans l'assiette des Français ce que l'on ne veut pas voir produire en France pour des raisons sanitaires. Où en sommes-nous, monsieur le ministre ? Pourquoi cette interdiction n'est-elle pas respectée ? n'est-elle pas respectée ? Qu'attendons-nous pour défendre nos agriculteurs ? La parole

de la demande. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la passion qui a animé l'ensemble des discours entendus cet après-midi constitue la preuve de l'importance du débat que nous venons d'avoir. Les tendances de fond qui bouleversent notre agriculture justifiaient un rapport tirant rapport tirant la sonnette d'alarme. Permettez-moi de remercier l'ensemble du groupe d'études Agriculture et alimentation du Sénat et son président, Laurent Duplomb, pour avoir relevé ce défi. Ce cri d'alarme a bien été entendu dans campagnes : pas un déplacement, pas un échange avec les agriculteurs sur le terrain sans que ce rapport soit mentionné. Il traduit, en réalité, une inquiétude profonde du monde agricole. Edgard Pisani- permettez-moi de regarder dans le rétroviseur, monsieur le ministre ! -, qui fut ministre de l'agriculture sous Charles de Gaulle, aurait-il pu imaginer que la France ne serait plus le premier exportateur agricole européen ? Christian Bonnet, sous Valéry Giscard d'Estaing, Michel Rocard, pendant les septennats de François Mitterrand, auraient-ils pu seulement croire que la France connaîtrait un déficit commercial agricole avec ses voisins européens ? Quand Jacques Chirac nous invitait à manger des pommes, la France n'importait pas, comme c'est le cas aujourd'hui, la moitié de ses fruits et légumes ! Cette dégradation rapide de nos positions agricoles sur les marchés mondiaux est aujourd'hui une réalité. C'est un drame pour nos agriculteurs bien sûr, sûr, qui- il faut le rappeler -tirent 25 % de leur revenu des exportations françaises. C'est d'ailleurs, peut-être, l'un des malentendus de la loi Égalim résoudre le problème du revenu de l'agriculteur en ciblant uniquement les ventes opérées par la grande distribution, c'est un peu court, comme aurait dit Cyrano ! Notre agriculture a besoin d'excellence et de compétitivité pour exporter. Plus largement, cette dégradation est surtout dommageable pour la France et contradictoire avec les demandes sociétales. Comment peut-on assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens alors même que nous importons dont- je le confirme -nous ne pouvons contrôler avec certitude la conformité non pas aux normes de qualité mais à nos normes de production ? Comment peut-on s'engager résolument en faveur d'une politique environnementale ambitieuse et se satisfaire de l'explosion du transport par cargo de denrées traitées parfois avec des molécules non autorisées en France ? À l'heure de conclure ce débat, je me félicite que nous partagions tous, quelles que soient nos étiquettes politiques, ces inquiétudes. Monsieur le ministre, vous êtes conscient de la situation et je vous remercie de vous être plié à cet exercice en répondant à nos questions si diverses. Toutefois, il faut que paroles et actes convergent. Malgré la sympathie que vous inspirez, je voudrais rappeler quelques éléments. Avec la signature à marche forcée, certes commencée sous d'autres mandats, l'agriculture française est à chaque fois la variable d'ajustement de l'Union européenne, vous allez accroître la part des importations dans la consommation des Français. Le CETA pose problème, non pas en raison de la qualité des produits que nous allons engendre une concurrence des modèles de production et une incohérence entre ce que nous demandons à nos agriculteurs et ce que nous acceptons des agriculteurs canadiens. Mais ce n'est pas tout ! Avec ce qui s'apparente à une nouvelle renationalisation de la PAC, vous allez également accentuer les concurrences déloyales au sein même de l'Union européenne. Avec la réduction du budget de la PAC à un niveau historiquement bas, vous semblez considérer que l'indépendance alimentaire de la France n'est pas suffisamment stratégique, alors même que les autres grands États ont augmenté leur budget agricole ces dernières années. Monsieur le ministre, nous ne pouvons plus affaiblir ni le revenu des agriculteurs ni leur capacité d'investissement. Il est urgent de réagir en favorisant les exportations- c'est une voie -, et donc en érigeant la compétitivité de notre agriculture au rang de priorité nationale. Nous sommes un grand pays agricole et le moment que nous vivons est stratégique, mes chers collègues. L'agriculture est à la convergence des grands défis auxquels nous devons collectivement faire face.

durable. Dans tous ces domaines, nous pouvons avoir une agriculture exportatrice de nos produits et de nos savoir-faire. Très bien ! Enfin, elle répond aux enjeux de fracture territoriale qui sont au coeur des problématiques locales de notre La meilleure façon de réaliser ses rêves, disait Paul Éluard, est de se réveiller. Alors, mes chers collègues, monsieur le ministre, collectivement, réveillons-nous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

la proposition de loi qui est examinée aujourd'hui a fait l'objet d'une procédure de législation en commission, la LEC. Dans le cas de cette proposition de loi, la LEC a montré qu'elle avait toute son utilité, non seulement pour traiter de sujets techniques, mais aussi pour permettre d'accélérer l'examen de textes très attendus. En effet, si ce texte peut, à première vue, sembler de l'ordre de l'ajustement technique, il est, en réalité, tout le contraire : il porte sur un sujet qui touche au quotidien des élus locaux, sur une difficulté à laquelle il est urgent d'apporter une solution. Ce sujet, c'est celui du poids administratif et financier de l'élaboration des documents locaux de planification. Nous connaissons bien les contraintes qui s'appliquent aux élus locaux. La proposition de loi de notre collègue Serge Babary traite du cas particulier des règlements locaux de publicité, les RLP : ce document de planification locale, similaire au plan local d'urbanisme, PLU, vise à réglementer les affichages publicitaires des villes, en durcissant ou assouplissant le droit commun national. Ce n'est pas la première fois que ce sujet des règlements locaux de publicité intercommunaux arrive devant notre assemblée. Il s'agit d'une demande exprimée de longue date par les communes et les intercommunalités. En effet, les élus locaux pâtissent des lourdes conséquences d'une articulation manquée entre trois lois successives

Ces trois lois, adoptées en moins de sept ans, témoignent de l'instabilité juridique qui touche les compétences locales et les documents de planification. intercommunale, doivent s'adapter très vite aux évolutions successives, au prix de délais d'élaboration allongés et de dépenses supplémentaires. Depuis la création des RLP, c'étaient principalement les communes qui étaient compétentes pour les élaborer. Mais depuis la loi ALUR, qui a organisé le transfert de la compétence de PLU et donc de RLP aux intercommunalités, les EPCI ont dû se saisir de cette nouvelle compétence. Or il faut en moyenne deux à trois ans pour élaborer un RLP intercommunal, alors que certains EPCI ont acquis cette compétence il y a à peine un an. En conséquence de ces évolutions rapides, il existe aujourd'hui non moins de quatre types de règlements locaux de publicité sur le territoire. À peine 5 % des RLP existants en France sont des RLP intercommunaux

Une contrainte supplémentaire vient encore compliquer la tâche des intercommunalités : pour inciter à l'élaboration de RLP conformes, la loi a prévu la caducité de tous les RLP de première génération au 14 juillet 2020. C'est demain ! Dans moins de dix mois, ce sont donc 1 211 documents locaux qui pourraient tout bonnement disparaître. Imaginez l'ampleur des conséquences pour les communes concernées ! Je vous en donnerai trois exemples. Premièrement, le règlement national de base s'appliquera au lieu des réglementations locales. Les maires risquent de voir fleurir des milliers d'affichages publicitaires sauvages, sans moyen de s'y opposer. Deuxièmement, le pouvoir de police de la publicité sera transféré au préfet, alors qu'il est dans les mains du maire sous le régime du RLP. Ce serait un dessaisissement des communes. Troisièmement, enfin, les collectivités perdraient les recettes liées au mobilier urbain et à la publicité dans les villes. Pour la seule métropole d'Aix-Marseille-Provence, cela représenterait une perte de 11 millions d'euros par an. L'autre problème auquel s'attaque la proposition de loi est le manque d'articulation entre les procédures applicables aux PLU et aux RLP. Alors que dans la plupart des cas, ce sont bien les mêmes EPCI qui élaborent ces deux documents, parfois simultanément, les procédures applicables n'ont pas été harmonisées. Par exemple, les grands EPCI tels que les métropoles peuvent élaborer des PLU dits « infracommunautaires » à l'échelle de territoires. Ces possibilités ne sont pas expressément prévues dans le cas des RLP. Or de nombreuses collectivités ont déjà entrepris d'élaborer ou de réviser leurs documents selon ces nouvelles procédures. Vous mesurez bien, mes chers collègues, que les communes et intercommunalités font face à une double urgence : il faut, d'une part, sécuriser les documents de planification déjà élaborés ou en cours d'élaboration, et, d'autre part, permettre à ces procédures d'être menées à leur terme avant que la caducité généralisée ne les frappe.

malgré un consensus, les deux articles relatifs aux RLP ont été censurés par le Conseil constitutionnel en novembre 2018, qui les a considérés ». La présente proposition de loi offre une nouvelle chance de prévoir les assouplissements nécessaires. Elle apporte deux solutions. D'abord, le texte reporte de deux ans l'échéance de caducité des RLP, mais uniquement dans le cas où l'EPCI s'est déjà engagé dans l'élaboration d'un RLP intercommunal conforme. Ensuite, le texte valide les RLP des intercommunalités qui ont appliqué de bonne foi des procédures non prévues par la loi, et précise que les assouplissements de procédure valables pour les PLU intercommunaux sont aussi valables pour les RLP intercommunaux. La commission des affaires économiques soutient pleinement les mesures proposées par le texte. Ce sont là deux mesures de bon sens, très attendues par les intercommunalités et les communes qui se trouvent aujourd'hui dos au mur. Lors de l'examen dans le cadre de la LEC, la commission a enrichi la proposition de loi sur trois volets.

aux dates d'entrée en vigueur de dispositions relatives à la publicité, en les alignant avec l'échéance de caducité. Vous l'aurez compris, il ne faut pas prendre cette proposition de loi à la légère.

du Gouvernement, Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, Monsieur le président, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi examinée cet après-midi a, comme vous l'avez dit, madame la rapporteur, pour objet de sécuriser et de conforter la dynamique d'élaboration volontaire de règlements locaux de publicité intercommunaux afin d'adapter la réglementation nationale aux enjeux locaux. Cet enjeu est fondamental pour l'attractivité des territoires. L'équilibre n'est pas toujours facile à trouver entre les objectifs de développement économique de ces territoires

Cependant, ces articles ont été censurés par le Conseil constitutionnel, qui les a considérés comme des cavaliers législatifs. Comme l'a rappelé ma collègue Brune Poirson en commission la semaine passée, cette censure ne remet en cause ni la pertinence des dispositions ni leur opportunité. Jusqu'au Grenelle de l'environnement, les communes élaboraient leur règlement local de publicité selon une procédure du code de l'environnement. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II, a adossé la compétence en matière de RLP à la compétence en matière de plan local d'urbanisme.

a prévu le principe du transfert de ces compétences aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Conséquence de ces deux lois, la compétence des EPCI en matière de RLP a été généralisée, ce qui a fait émerger de nouvelles difficultés, que la présente proposition de loi entend résoudre. Premièrement, dans la mesure où les procédures des RLP sont calquées sur celles des PLU, toute élaboration ou évolution d'un RLP par un EPCI doit se faire sur la totalité du territoire de l'EPCI, sans dérogation possible. Or la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a permis l'élaboration de PLU infracommunautaires, ne couvrant pas l'intégralité de leur territoire,

En outre, cette situation engendre une forme d'insécurité juridique, car plusieurs EPCI ont déjà engagé l'élaboration de RLP infracommunautaires, en pensant que les aménagements de la loi du 27 janvier 2017 étaient suffisants. Deuxièmement, la loi Grenelle II a prévu que les anciens RLP, dits « de première génération », restaient valables jusqu'à leur révision, et pour une durée maximale de dix ans à compter de la publication de la loi. Ils seront donc caducs le 14 juillet 2020, ce qui constitue une échéance trop brève. En effet, de nombreux EPCI sont devenus compétents en matière de PLU et de RLP ou sont concernés par une création, une fusion ou une modification de leur périmètre. Il est donc nécessaire d'accorder un délai supplémentaire à la révision des règlements locaux de publicité, d'où la proposition de deux années supplémentaires pour les EPCI ayant prescrit l'élaboration d'un RLP intercommunal. En outre, plusieurs améliorations notables ont été adoptées en commission, sur proposition de Mme la rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement. Je pense aux EPT de la métropole du Grand Paris, qui ne disposent pas du statut d'EPCI à fiscalité propre, mais qui bénéficieront également du report de la caducité des RLP de première génération. Je pense ensuite à l'introduction d'un délai de deux ans pour permettre aux professionnels, après la caducité des RLP de première génération, de mettre en conformité avec la réglementation nationale leurs publicités, enseignes et préenseignes. à la coordination de la date d'entrée en vigueur d'une mesure de la loi du 7 juillet 2016, qui s'appuie sur la date de caducité des RLP de première génération, avec le report de cette date. Enfin, conformément à l'engagement pris par Brune Poirson en commission, je voudrais apporter la réponse du Gouvernement à une inquiétude exprimée sur les conséquences de l'adoption d'un RLP intercommunal en termes de pertes financières des communes au profit des intercommunalités : il n'y en aura pas,

De prime abord, cette proposition de loi semble ne procéder qu'à un simple ajustement réglementaire, mais tant s'en faut. En effet, les règlements locaux de publicité, similaires aux plans locaux d'urbanisme, permettent de réglementer les affichages publicitaires des villes. En la matière, ils donnent la possibilité au maire de définir les zones dans lesquelles les règles applicables dérogent au droit commun national, mais aussi de soumettre certains affichages à son autorisation. Cette compétence a donc un impact direct sur la qualité de notre cadre de vie, mais aussi sur l'environnement. Depuis sa création dans les années 1980, il revenait généralement aux communes d'élaborer les RLP. Cependant, une série de trois lois est venue remettre en cause cette compétence communale. portant engagement national pour l'environnement a lié RLP et PLU, puis la loi ALUR du 24 mars 2014, en transférant le PLU aux intercommunalités, a mécaniquement transféré la compétence des RLP aux EPCI. et à la citoyenneté de 2017. Ces modifications successives ont eu un impact important. D'une part, il y a eu multiplication des types de RLP, puisqu'il en existe désormais quatre : ceux adoptés sous l'ancien format par les communes et antérieurs à 2010, dits « de première génération ceux adoptés entre 2010 et 2011 dits « transitoires », ceux de deuxième génération adoptés par les communes selon le modèle imposé en 2010 ; et enfin les RLP intercommunaux adoptés par les EPCI depuis 2010. Cela fait beaucoup ! Dans les faits, il existe aujourd'hui 1 681 RLP, mais seulement 82 sont intercommunaux, alors que 72 % des RLP, soit 1 211, ne sont pas conformes puisque adoptés avant 2010. D'autre part, afin d'inciter à l'élaboration des règlements locaux de publicité intercommunaux, la loi de 2010 a organisé la caducité de tous les RLP de première génération au 14 juillet 2020, remettant en cause les 1 211 RLP existants. De fait, cela entraînerait l'application du règlement national de base, généralement moins protecteur, en lieu et place des réglementations locales. Cela ne sera pas sans conséquence, notamment sur la multiplication des affichages sauvages,

En outre, et ce n'est pas la moindre des conséquences, les recettes tirées du mobilier urbain et de la publicité dans les villes ne reviendraient plus aux collectivités. Face à cette situation, la proposition de loi vise à rendre applicables aux RLP les aménagements, la révision, la modification et la caducité des PLU par par la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017. L'article 1prévoit notamment de laisser la possibilité de déroger, dans certains cas, au principe posé par le code de l'environnement, selon lequel le RLP doit être élaboré sur l'ensemble du territoire de l'EPCI. Cette disposition sécuriserait les EPCI issus d'une fusion d'EPCI et leur éviterait de reprendre la procédure d'élaboration à zéro. Quant à l'article 2, il a trait

En la matière, il s'agit donc d'accorder à ces EPCI nouvellement compétents en matière de PLU un délai supplémentaire de deux ans pour transformer les RLP de première génération en RLP de deuxième génération. Reste que la question soulevée en commission des affaires économiques par notre collègue Martial Bourquin sur l'affectation du produit de la publicité dans le cadre de RLP intercommunaux est essentielle, et qu'elle demeure sans réponse. Il ne faudrait pas que les communes se retrouvent privées de ces finances indispensables notamment à l'activité des centres et centres-bourgs de nos villes. Si tel était le cas, cela signifierait la disparition, une nouvelle fois, de ressources dédiées aux communes, ce qui n'est pas acceptable.

défini par le code de l'environnement, est un outil communal et intercommunal de planification de l'affichage publicitaire. Il est destiné à réglementer, généralement dans un sens plus restrictif que le règlement national, la publicité, les enseignes et préenseignes, dans un but de protection du cadre de vie et des paysages, tout en assurant un équilibre avec le droit à l'expression et à la diffusion d'informations et d'idées. et d'idées. Ces espaces d'information n'ont pas pour unique raison d'être la publicité commerciale ; ils sont aussi un support important, voire essentiel, d'une information à caractère évènementiel, touchant à des domaines aussi divers que la culture, le patrimoine, les sports ou les manifestations festives. La préenseigne peut également être pertinente d'un point de vue environnemental, lorsqu'elle permet d'éviter la surcharge d'une panneautique publique ou, pis encore, le fléchage sauvage d'établissements commerciaux ce fléchage d'orientation, toujours nécessaire malgré les GPS, est particulièrement le fait des hôtels et des restaurants. Depuis 2010, l'EPCI, compétent en matière de plan local d'urbanisme, ou PLU, est également de plein droit compétent en matière de règlement local de publicité

et des tensions plus marquées entre les communes et leur EPCI. Quant à la chimère des économies d'échelle, elle est à nouveau mise en avant, alors que le risque est inverse ; il ne peut y avoir d'économies d'échelle que lorsqu'il y a partage de frais fixes. Or, dans ce cas, le coût d'élaboration porte essentiellement sur des frais plus ou moins proportionnels au nombre de communes et à la taille du territoire. Le règlement local de publicité est un outil qui peut, certes, reposer sur de grands principes, mais qui reste du « cousu main », pour s'adapter aux caractéristiques de chaque territoire. Quel intérêt absolu y aurait-il à harmoniser les règlements de publicité sur des EPCI « XXL », ayant des caractéristiques très différentes en matière topographique, d'habitat ou d'environnement naturel ? En l'état, quelque 60 % des règlements locaux de publicité élaborés avant 2010 deviendraient caducs en juillet 2020. Repousser cette date de deux ans me semble donc une proposition,

Doit-on faire un parallèle avec la taxe d'aménagement ?

La structure qui bénéficiera des recettes aura une approche différente du règlement local de publicité ; et, dans un sens comme dans l'autre, quelle que soit l'hypothèse retenue, on se trouve confronté à une sorte de conflit d'intérêts.

Malgré ces observations et ces critiques, le groupe du RDSE ne s'opposera pas à l'adoption de ce texte, dont l'objet principal est de proroger de deux ans la mise en oeuvre d'un dispositif prévu par des lois plus anciennes, datant des deux précédents quinquennats. La parole est à M. François

Cette proposition de loi visant à encourager l'adoption de règlements locaux de publicité intercommunaux répond à une problématique très importante pour nos collectivités. C'est la raison pour laquelle je tiens à remercier nos collègues Serge Babary, auteur de la proposition de loi, et Dominique Estrosi Sassone, rapporteur, pour leurs travaux. Cette proposition de loi, nous l'avons en réalité déjà examinée, et même votée à l'unanimité. En effet, elle reprend les articles 52 et 53 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN. Le Conseil constitutionnel a malheureusement censuré ces articles, considérant qu'ils n'avaient pas de lien avec le texte initial. Il ne s'agit pas simplement d'un détail technique ou d'une mesure de coordination ; il s'agit d'une mesure essentielle, attendue par près de 1 200 communes concernées. Ce texte adapte la réglementation nationale aux enjeux locaux, en matière d'élaboration volontaire des règlements locaux de publicité intercommunaux.

de textes qui ont transformé le dispositif. Aujourd'hui, ce dernier est confronté à un vide juridique, qui rend difficile son application locale. Des EPCI se retrouvent même dans des situations d'insécurité juridique, entraînant une paralysie des procédures en cours. Le groupe La République En Marche votera donc en faveur de cette proposition de loi, très attendue par nos collectivités. Madame la secrétaire d'État, vous avez répondu par avance aux questions soulevées par certains d'entre nous. groupe est également en accord avec les apports de la commission, pour donner un délai de deux ans de mise en conformité. Madame la secrétaire d'État, nous connaissons votre engagement pour les collectivités ; vous avez toute notre confiance pour que cette proposition de loi soit adoptée dans les meilleurs délais. La parole

vote. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, pour la énième fois- il faut croire que cela va devenir une habitude -, nous revenons, par le biais d'une proposition de loi, sur des mesures définies comme cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel.

Un tel constat ne peut que nous inquiéter quant aux prérogatives des parlementaires et à leur capacité réelle à enrichir les projets de loi soumis par le Gouvernement, à l'heure où vont bientôt s'ouvrir les débats sur la révision constitutionnelle. Le message envoyé et la place du législateur dans le débat public demeurent préoccupants. Pour en revenir au texte que nous étudions aujourd'hui, rappelons, s'il en était besoin, le rôle fondamental que jouent les PLU et les règlements locaux de publicité dans la politique d'aménagement local. Ils permettent de réglementer l'utilisation de l'espace et, donc, la cohabitation d'intérêts divergents. Il semble donc cohérent que ces deux documents de planification et de réglementation, qui participent aux mêmes exigences de maîtrise urbaine, puissent être conduits, dans leur réalisation, au même échelon. Dans ce contexte, nous sommes convaincus que les élus doivent disposer d'outils efficaces leur permettant de définir le cadre du développement de la publicité sur leur territoire. S'il faut respecter la liberté d'expression et la liberté d'entreprendre, il est également nécessaire de prévoir des garde-fous contre une publicité intempestive, qui défigure le plus souvent les entrées de ville.

via ces règlements, la protection des secteurs d'intérêt patrimonial, architectural ou paysager, ainsi que la qualité du cadre de vie, tout en laissant la souplesse nécessaire à la prise en compte de situations particulières et de circonstances locales. Nous considérons que l'échelon intercommunal peut et doit produire des effets positifs, comme la mutualisation des moyens, la lutte contre les effets de frontière grâce à l'homogénéisation des pratiques, et l'intégration de la gestion de la publicité à un projet de territoire porté à l'échelon intercommunal.

Afin d'accompagner celles-ci, nous soutenons, depuis le début, l'impérieuse nécessité d'ériger uniquement des intercommunalités choisies, et fondées sur un projet commun, permettant ainsi de respecter la volonté des communes, au regard du caractère très engageant et fondateur de ces documents, qui traduisent très directement les politiques municipales. Qu'il s'agisse de la définition du PLU ou de celle du RLP, nous considérons que ces compétences doivent être librement transférées aux intercommunalités.

plus de temps aux intercommunalités pour produire un règlement local de publicité, conformément à la loi portant engagement pour l'environnement, en repoussant l'échéance de 2020, année électorale, à 2022. Cela paraît être un bon dispositif, qui incite les élus à s'engager. Il est nécessaire d'accorder un délai supplémentaire de deux ans, car, je l'ai dit en commission, un cadre assoupli évitera que les équipes nouvellement élues en 2020 aient à mettre en oeuvre un RLP

Merci

La publicité par voie d'affichage est un outil de communication utile, qui doit bénéficier à tous ; c'est, avant tout, l'un des modes d'exercice de la liberté d'information, et la publicité contribue bien évidemment à faire vivre le tissu économique des collectivités territoriales. À titre personnel, je suis tout à fait favorable aux panneaux qui relaient les informations du service public, mais je suis résolument contre les panneaux commerciaux, ceux qui annoncent les grandes surfaces ou les promotions sur les meubles ; j'en passe, et des meilleures. Il nous faut davantage informer sur les évènements culturels ou sportifs, sur les foires-expositions, sur notre patrimoine, sur les zones économiques des collectivités. Il nous faut faire connaître les évènements organisés par l'ensemble des collectivités territoriales, mais aussi par les associations ; ce sont ces manifestations qui font vivre

La France est un pays riche de ses villes, de ses villages, de ses campagnes, de son patrimoine. Nous devons communiquer sur ses atouts. nous sommes tous attachés au développement de nos territoires, la publicité ne doit pas non plus défigurer nos villes ni nos paysages ; pour cela, nous avons les éoliennes. La réglementation et plus encore la planification sont indispensables et doivent être adaptées aux particularités locales. L'excellente proposition de loi de notre collègue Babary clarifie le droit existant et repousse de deux ans la caducité des règlements locaux de publicité. Ces documents sont techniques et complexes. Ils demandent du temps- parfois quatre ou cinq ans -et de l'argent ; les deux manquent aux collectivités. J'espère que l'alignement de la procédure d'élaboration des règlements locaux de publicité sur celle des plans locaux d'urbanisme permettra de régulariser les procédures engagées, avant la loi NOTRe, par les établissements particulièrement diligents. À défaut, ces établissements devront recommencer leur procédure, qui représentera évidemment un coût et du temps. La commission a complété utilement le texte. Si rien n'est fait, plus de mille EPCI EPCI se verront appliquer, au 14 juillet 2020, le règlement national de publicité, moins protecteur et moins adapté. Ce règlement prévoit surtout- c'est essentiel pour les collectivités -que la police de l'affichage est exercée par le préfet et non plus par le maire, et que les collectivités ne perçoivent plus les taxes afférentes au mobilier urbain. À l'heure où l'on demande plus de proximité, cela n'est évidemment pas souhaitable, et cela n'est financièrement pas envisageable pour les collectivités.

la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, et qui a été étudiée selon la procédure de législation en commission, peut sembler technique. Néanmoins, elle est essentielle pour les élus locaux, qui attendent de nous des décisions clarifiant le droit, simplifiant les règles d'urbanisme et encourageant l'amélioration du cadre de vie. La situation actuelle en matière de règlements locaux de publicité intercommunaux- l'examen de cette proposition de loi le rappelle -résulte de l'empilement de lois successives, votées majorité après majorité, souvent rapidement, généralement pour satisfaire de grands enjeux en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, mais rarement pour simplifier la vie des élus locaux. Pas moins de trois lois successives ont touché aux règles d'urbanisme. Ces textes, parfois contradictoires, ont surtout contraint les communes et les intercommunalités à s'adapter, comme elles le pouvaient, dans des délais difficiles à tenir. La question des RLP, traitée aujourd'hui, en est une conséquence et une illustration. Nous sommes arrivés à un état d'insécurité juridique très fort, en raison de délais incohérents ou intenables, eu égard aux procédures d'élaboration de ce type de documents. Si l'on ne peut que souscrire, sur le fond, à ce texte, celui-ci doit nous rendre collectivement- tant le Gouvernement que le Parlement - conscients des conséquences de nos décisions. Les élus locaux sont épuisés par les changements de règles, ils sont inquiets pour l'avenir et ils se sentent exposés par les responsabilités qui pèsent sur eux.

fait surtout pour la préservation des paysages, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des entrées de ville et de l'harmonie de nos communes. Vous connaissez tous ici mon attachement aux questions relatives au patrimoine et à sa protection. Nous devons aider les élus locaux à acquérir des outils qui leur permettent d'assurer ces objectifs essentiels. On parle beaucoup d'environnement dans l'actualité, et le sujet que nous traitons ici en fait pleinement partie, au titre de la pollution visuelle et de la protection du patrimoine. Dans une vie antérieure, lorsque je présidais le parc naturel régional de la Montagne de Reims, j'ai participé à la création et à l'élaboration d'une charte et d'un règlement pour les publicités, enseignes et préenseignes, afin d'améliorer la qualité des paysages de nos communes. Rapidement, ce travail a été une référence pour les autres parcs régionaux, sur laquelle ceux-ci ont pu s'appuyer pour élaborer leur règlement de publicité. Les publicités, enseignes et préenseignes, sont soumises à une réglementation protectrice de l'environnement et du cadre de vie. Leur installation doit être conforme à des conditions de densité et de format, et faire l'objet de déclarations ou d'autorisations préalables en mairie ou en préfecture. Le règlement local de publicité, qu'il soit communal ou intercommunal, est un acte volontariste, destiné à encadrer ces conditions d'installation, et les adapter au territoire communal ou intercommunal. En zone rurale, il faut souvent trouver un équilibre entre protection visuelle et désenclavement, donc attractivité économique ou commerciale. Ainsi, la question des enseignes et préenseignes, annonçant les restaurants traditionnels de nos communes, pose souvent question. Un équilibre a été retrouvé ; il permet de mettre en avant les activités liées également aux produits locaux. C'est un bon compromis, qu'il ne faudrait pas déstabiliser. Les RLP sont un bon outil, à condition de laisser les élus s'en emparer. Chaque collectivité peut d'ailleurs se faire conseiller, notamment pour aménager ses entrées de ville ; je crois que c'est essentiel. Après avoir salué le travail toujours efficace de notre rapporteur,

nous examinons aujourd'hui la proposition de loi que j'ai déposée avec plusieurs de mes collègues, dont Mme Primas, présidente de la commission des affaires économiques, Mme Estrosi Sassone, rapporteur du texte, et Mme Lamure. Je remercie celles-ci de leur soutien ; cette proposition de loi est attendue par de très nombreux élus locaux.

en tant que cavaliers législatifs. C'est donc non pas le fond, mais le choix du support qui a été censuré par le juge constitutionnel. Les débats ayant déjà eu lieu, et un consensus ayant été trouvé, il est important d'inscrire ces dispositions dans le code de l'environnement.

Il est destiné à réglementer la publicité, les enseignes et préenseignes, dans un but de protection du cadre de vie et des paysages, tout en assurant l'équilibre avec le droit à l'expression et à la diffusion d'informations et d'idées. Il permet d'adapter localement le règlement national de la publicité.

Pour plus de simplicité, cette loi a également prévu que ce règlement serait élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures définies par le code de l'urbanisme pour l'élaboration, la révision ou la modification des PLU. Par la suite, la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR a généralisé le transfert automatique de la compétence relative au PLU aux intercommunalités, et donc, par ricochet, de celle de l'élaboration du règlement local de publicité. Ce transfert automatique a requis plusieurs ajustements relatifs à l'élaboration et à la modification des PLU, qui ont été mis en oeuvre par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Ces aménagements n'ont malheureusement pas été explicitement étendus aux règlements locaux de publicité. Aussi, l'article 1 de la présente proposition de loi a pour objet de sécuriser juridiquement l'élaboration des RLP intercommunaux, en leur rendant applicables ces aménagements. L'article 2, quant à lui, a pour objet d'aménager l'échéance de caducité des règlements locaux de publicité, en la repoussant de deux ans. En effet, l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement, institué par la loi Grenelle II, prévoit que les anciens RLP seront caducs au 14 juillet 2020. Cette échéance, arrêtée en 2010, ne tient évidemment aucun compte du transfert de la compétence relative au PLU aux intercommunalités, transfert qui a été voté en 2014. Compte tenu du coût et de la complexité de l'élaboration d'un RLP intercommunal, cette échéance ne pourra être tenue par les EPCI nouvellement compétents en matière de PLU. En effet, selon l'Union de la publicité extérieure, sur les 1 258 établissements publics intercommunaux, seuls 125 ont lancé la procédure, et, sur les 13 établissements qui ont adopté leur nouveau règlement, 5 seulement comptaient plus de 100 000 habitants. Ces chiffres montrent à eux seuls l'urgence de la situation. Si aucun règlement local n'est adopté avant la date butoir de juillet 2020, c'est le règlement national qui s'appliquera. Or il est essentiel de permettre aux acteurs locaux d'établir une politique publique de l'affichage, et de définir des règles adaptées à leurs territoires. Il s'agit, avant tout, d'éviter l'application du règlement national de publicité et de s'assurer de la proximité de la règle établie. Il s'agit ainsi d'éviter que le maire ne soit dessaisi, au profit du préfet, de son pouvoir de police de la publicité, mais aussi d'éviter que les collectivités ne perdent les recettes liées au mobilier urbain et à la publicité. L'article 2 modifie donc cette échéance en instaurant un délai supplémentaire de deux ans. l'initiative de Mme le rapporteur, la commission a étendu cette disposition aux établissements publics territoriaux du Grand Paris, et a ajouté deux articles. Le premier- l'article 3 de la proposition de loi -offre un temps d'adaptation et de sécurité juridique. En l'absence d'adoption d'un RLP intercommunal, les collectivités auront deux ans supplémentaires pour mettre en conformité l'affichage avec le règlement national. Le second- l'article 4 du texte -coordonne l'entrée en vigueur des RLP intercommunaux avec la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

Enfin, je retiens l'engagement du Gouvernement que cette proposition de loi soit rapidement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. J'y insiste, il est impératif que cette proposition de loi puisse être votée et promulguée avant l'été prochain. Personne ne

La séance est suspendue.

Le Gouvernement reconnaît que certaines formes d'actions militantes contreviennent au libre exercice d'activités autorisées par la loi et que ce sujet mérite d'être examiné par le Parlement.

Pour revenir à la chasse, cet été, de nombreuses fédérations de chasseurs ont vu leur siège attaqué ou incendié. Tous ces exemples, que l'on pourrait multiplier à l'envi, montrent que notre société est malade.

Il était nécessaire de faire évoluer l'arsenal répressif pour l'adapter à ces nouvelles formes de contestation que constituent l'entrave ou l'obstruction passive, véhiculées sur les réseaux sociaux par des activistes souvent non solvables, pour qui la sanction contraventionnelle reste sans effet. Il était donc impératif d'adapter l'article 431-1 du code pénal à cette évolution relativement récente, pour rendre la sanction plus universelle, avec comme principe de base le fait que chacun puisse défendre ses idées dans un cadre légal par la communication, la persuasion, voire des propositions faites au législateur, mais pas par la force et la violence. C'est du simple bon sens, qu'il faut traduire en droit.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons cet après-midi la proposition de loi déposée par notre collègue Jean-Noël Cardoux tendant à réprimer les entraves à l'exercice des libertés, ainsi qu'à la tenue des évènements et à l'exercice d'activités autorisées par la loi. Ce texte vise à apporter une réponse plus ferme et plus efficace à deux types d'infractions qui ont eu tendance à se multiplier ces dernières années et qui, à certains égards, relèvent d'un phénomène de société : les violences, les menaces et les dégradations dirigées contre des boucheries, des abattoirs ou des élevages, en général au nom d'une conception très singulière et exclusive de la cause animale les entraves à la chasse, qui se produisent régulièrement dans nos forêts domaniales. Ces actions sont le fait de groupes ou d'individus radicaux issus en général de mouvements animalistes, antispécistes ou véganes, apparus voilà une trentaine d'années, mais dont certains modes d'action ont pris une forme violente plus récemment. Au cours de la seule année 2018, la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs a ainsi recensé une cinquantaine d'attaques, sous des formes diverses et variées : vitrines brisées, murs tagués, faux sang répandu dans les boutiques, bouchers ou clients menacés ou insultés. Certains évènements, comme des attaques contre les agriculteurs, ont pu prendre un tour plus dramatique. Je pense en particulier à l'incendie de bâtiments d'élevage, il y a encore dix jours, dans l'Orne, où un jeune exploitant agricole a vu, en pleine nuit, ses trois bâtiments d'élevage détruits par le feu.

Je pense aussi à l'incendie volontaire, voilà un an, d'un l'abattoir dans le département de l'Ain : s'il n'a heureusement pas fait de victimes, cet incendie criminel a mis au chômage technique près de quatre-vingts

Au demeurant, est-il nécessaire de réaffirmer ici que la chasse, acquis historique s'il en est, reste un loisir apprécié du plus grand nombre, avec près de 1 million de pratiquants et détenteurs de permis de chasse de notre pays ? Je rappelle que les entraves à la chasse sont aujourd'hui réprimées par une simple contravention de cinquième classe, soit une amende de 1 500 euros au maximum, ce qui, manifestement, n'est plus assez dissuasif. Plus généralement, il y va du respect de l'une de nos libertés les plus fondamentales. Je crois que nous vivons, en France, dans un pays de libertés, où toutes les opinions peuvent s'exprimer dignement et être défendues librement. Aussi, les militants animalistes ont tout loisir de s'opposer, par exemple, à la consommation de la viande, à la considérer comme impure, de s'opposer à la chasse, à la corrida ou encore à la présence d'animaux sauvages dans les cirques. C'est leur droit, mais c'est parce que notre démocratie leur permet de s'exprimer librement qu'elle ne peut admettre que l'on cherche à imposer son opinion par la force. C'est même le propre de notre État de droit que nul ne saurait imposer ses opinions par la violence ou l'intimidation. Je rappelle également que, face à la multiplication de ces incidents, le ministre de l'intérieur a demandé aux préfets de région de prendre contact avec les représentants des professions concernées pour des échanges réguliers et pour leur fournir une protection si nécessaire.

La chancellerie a, de son côté, invité les procureurs à faire preuve de fermeté contre ceux qui attaquent des boucheries ou qui s'introduisent dans des élevages, en apportant une réponse systématique à ces actes, mais aussi en tentant de prévenir les débordements. les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent aujourd'hui aller plus loin, en modifiant l'article 431-1 du code pénal, leur objectif étant de réaffirmer un principe général selon lequel toutes les activités qui ne sont pas interdites doivent pouvoir être exercées librement, sans que certains tentent d'y apporter des entraves. L'article 431-1 du code pénal punit ainsi d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver, par une action concertée et au moyen de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, d'association, de réunion et de manifestation ou encore de la liberté du travail. Il punit des mêmes peines les entraves au bon déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'une collectivité territoriale. De même, les peines encourues sont alourdies- trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende -lorsque l'entrave a pris la forme de coups, de violences, de voies de fait, de destructions ou de dégradations. La proposition de loi tend à apporter deux modifications à cet article, afin d'en élargir le champ d'application. Tout d'abord, il est proposé de préciser que l'entrave est réalisée « par tous moyens », de manière à pouvoir sanctionner toutes les entraves, quelle qu'en soit la forme. Ensuite, le texte prévoit de sanctionner le fait d'empêcher la tenue de tout évènement ou l'exercice de toute activité autorisée par la loi. Je rappelle que la proposition avait déjà été inscrite à l'ordre du jour de notre

Le Gouvernement, depuis lors, a fait part de son intérêt pour ce texte, à l'occasion de l'examen du projet de loi portant création de l'Office français pour la biodiversité, au mois d'avril dernier. répondant à un amendement de notre collègue Jean-Noël Cardoux, qui tendait à créer un délit d'entrave à la chasse, la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon avait souhaité une inscription rapide de la proposition de loi à l'ordre du jour des assemblées, afin que la question de la chasse puisse être abordée

Cette prise de position ne traduit cependant pas un désaccord avec les objectifs des auteurs de la proposition ; elle est plutôt la conséquence d'interrogations de nature juridique. un certain nombre de nos collègues se sont inquiétés de la formulation d'un principe de portée très générale, qui pourrait poser une difficulté au regard du principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi pénale. En effet, je rappelle qu'une infraction doit être définie en des termes suffisamment précis pour que la peine soit prévisible et afin d'éviter ainsi tout risque d'arbitraire. plusieurs membres de la commission se sont demandé s'il était nécessaire de légiférer de nouveau et si les dispositions en vigueur ne permettaient pas déjà de réprimer les comportements visés. Il est vrai que certaines qualifications pénales peuvent être retenues, en fonction de la nature des actes qui ont été commis, pour poursuivre les infractions commises par des groupes animalistes. non exhaustive, les qualifications suivantes : menaces, violences, violation de domicile, incendie criminel, dégradation de biens privés en réunion ou encore provocation à un crime ou à un délit. Ce rappel étant fait, monsieur le secrétaire d'État, il nous semble toutefois que le droit pénal ne permet pas d'appréhender efficacement certaines situations d'entrave situées aux interstices, dans lesquelles les individus font obstacle par leur corps à l'exercice d'une activité, sans que leur action s'accompagne pour autant de menaces ou de violences. Nous croyons également utile d'envoyer un message politique fort, afin d'inviter les pouvoirs publics à la fermeté et de rappeler les règles qui doivent régir la vie collective ou la vie en société. C'est pourquoi j'ai travaillé avec l'auteur de la proposition de loi et avec d'autres collègues de l'Union Centriste à une nouvelle rédaction, à même d'apporter plus de précisions tout en restant fidèle aux objectifs du texte. La commission a ainsi adopté l'amendement de réécriture globale déposé par notre collègue Jean-Paul Prince, comme j'aurai l'occasion de vous l'expliquer suite de la discussion. En conclusion, mes chers collègues, je tiens à souligner que cette proposition de loi répond à une attente très forte de nos concitoyens, qui sont de plus en plus exaspérés par certains comportements contraires au pacte républicain. Il s'agit en fait d'un texte de liberté, qui vise à renouer avec un principe essentiel énoncé à l'article V de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ». La parole

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, notre droit est protecteur des libertés. C'est un fondement de notre démocratie, et nous y sommes tout particulièrement attachés. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui part d'une intention louable : celle de renforcer la protection des libertés individuelles et de prendre en compte l'évolution de plus en plus violente des mouvements de contestation. En particulier, cette proposition de loi vise les entraves à la chasse et les violences répétées menées contre certaines professions- j'y reviendrai. Avant toute chose, je tiens bien sûr, au nom du Gouvernement, à condamner extrêmement fermement les violences de tout type. La liberté de contester et de s'opposer est un droit fondamental, la violence, elle n'est pas excusable. Le Président de la République et le Premier ministre ont fait part, à l'issue du grand débat national, de leur volonté qu'un plan contre les violences soit mis en place. Avec le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner, nous sommes pleinement mobilisés contre la banalisation de la violence et je veux vous dire notre détermination. Aussi, le texte que nous examinons aujourd'hui prévoit d'étendre les dispositions de l'article 431-1 du code pénal sur le délit d'entrave, de deux manières par la suppression de l'exigence de menaces pour une entrave portant sur la liberté d'expression, de travail, d'association ou de manifestation- l'expression l'expression « par des menaces » serait ainsi remplacée par l'expression « par tous moyens », beaucoup plus générale - ; de l'autre, par la création d'une cinquième forme d'entrave, réprimant « le fait d'empêcher la tenue de tout évènement ou l'exercice de toute activité autorisée par la loi ».

La rédaction retenue pour une nouvelle cinquième forme d'entrave demeure extrêmement large et imprécise. Les infractions ne sont pas suffisamment caractérisées. Leur spectre d'application est trop large, ce qui pourrait nécessairement comporter une part d'arbitraire dangereuse pour l'équilibre des droits. De ce fait, il est probable que de telles dispositions soient censurées par le Conseil constitutionnel. Si cet obstacle est suffisant justifier la position du Gouvernement, les modifications apportées par la proposition de loi ne semblent du reste pas nécessaires au regard des objectifs du texte. En effet, l'exposé des motifs fait état d'un certain nombre de cas où la proposition de loi s'appliquerait. Je ne vais pas en faire la liste, mais on compte notamment les blocus empêchant les spectateurs d'assister à des spectacles, les actions empêchant certains commerçants de réaliser leurs ventes ou encore, comme cela a été mentionné dans les travaux réalisés autour de la proposition de loi, pour entraver la pratique de la chasse. Or il apparaît que toutes ces entraves sont d'ores et déjà couvertes par l'article 431-1 du code pénal ou sont sous le coup d'incriminations spécifiques. Pour ne citer qu'un exemple, l'article R. 428-12-1 du code de l'environnement prévoit une sanction en cas d'obstruction à des actes de chasse. De fait, la proposition de loi ne paraît pas utile, et sa constitutionnalité est à nouveau questionnable au nom du principe de nécessité des peines.

à ce phénomène, afin d'améliorer son action et de mieux travailler en coordination avec les services de renseignement, qui se mobilisent de plus en plus sur ces thématiques. Comme je le disais au début de mon intervention, nous ne tolérons aucune violence et nous n'acceptons pas phénomène puisse toucher gratuitement nos éleveurs, nos artisans ou nos chasseurs. Nous les soutenons et nous continuerons à chercher avec eux, avec les forces de l'ordre, avec les services de renseignement et les parquets, les meilleurs moyens pour les protéger.

elles interviennent immédiatement sur les lieux d'infraction, renforcées en tant que de besoin par des unités spécialisées dans le maintien de l'ordre. Elles conduisent également des investigations minutieuses, qui permettent d'identifier les auteurs de ces exactions et de les faire condamner.

sur les lieux, en plus des renforts en unités locales, pour sécuriser le site. Le contrôle d'un certain nombre de militants a été opéré et des investigations judiciaires ont été lancées, y compris avec nos partenaires étrangers. Je pense également- il est très important que vous le notiez -à l'interpellation en flagrant délit de sept militants qui tentaient d'incendier un abattoir sur la commune de Jossigny, action qui a pu être entravée grâce à l'action de nos services de gendarmerie : dix individus sont aujourd'hui mis en examen sous douze chefs d'inculpation et sont placés sous contrôle judiciaire. Dans le département du Nord, face à la multiplication d'actions de vandalisme qui ont été perpétrées par des militants radicaux, notamment à l'encontre de boucheries, les investigations ont abouti à plusieurs opérations judiciaires au cours desquelles une dizaine d'individus ont été interpellés

notamment dans le cadre de la chasse à courre. Face aux situations les plus sensibles- je pense aux départements de la Vendée ou de l'Oise -, la gendarmerie met systématiquement en place un large dispositif de sécurité pendant la période de chasse, notamment des patrouilles à cheval.

et des activités symboliques de la filière viande, comme les parties de chasse, les élevages bovins ou autres, les abattoirs et les boucheries. Le respect de l'autorité de la loi et des droits qu'elle consacre a toujours été défendu par le groupe RDSE. Nous condamnons donc toujours les débordements que l'on observe- boucheries vandalisées et d'abattoirs incendiés. Ce sont des atteintes aux biens défendues par le code pénal, qui méritent d'être poursuivies et sanctionnées. Elles le sont d'ailleurs déjà, dans les conditions que permet notre système carcéral à bout de souffle, une réalité administrative qui n'échappe à personne ici. Notre rapporteur nous a indiqué ce matin avoir reçu la confirmation de la Chancellerie que des instructions avaient été transmises, afin de mieux sanctionner les entraves lorsqu'elles entrent dans le champ de l'article 431-1, ainsi que les intrusions, les vols et violences avérés. C'est donc la preuve que notre collègue Jean-Noël Cardoux a été entendu et que le droit en vigueur permet déjà, à lui seul, à condition d'être mieux appliqué, de protéger les intérêts des professionnels concernés. Conformément aux arguments juridiques de clarté de la loi pénale et de proportionnalité qui ont été avancés en commission des lois, nous nous inquiétons des atteintes aux libertés d'expression et de manifestation qui pourraient en résulter, y compris d'ailleurs pour les professions que la proposition de loi vise à protéger

». En outre, la notion de délit d'entrave serait étendue, cette fois aux actions visant à « empêcher la tenue de tout évènement ou l'exercice de toute activité autorisée par la loi La mention « par tous moyens » pourrait donner lieu à des interprétations plus extensives dans les juridictions, alors que la rédaction actuelle bénéficie d'une interprétation stable et restrictive. En commission, nos voix ont été à l'unisson pour s'opposer à l'adoption de dispositions pénales manquant de caractérisation, donc de clarté. Dans la même veine, le principe de proportionnalité des peines, constitutionnellement garanti, s'oppose à ce que soient sanctionnées de la même manière des entraves à l'exercice des libertés fondamentales et celles d'activités de loisirs ou encore toute autre activité, simplement parce que celles-ci seraient « autorisée[s] par la loi ». Par ailleurs, lorsque l'article 431-1 a été inséré dans le code pénal, l'objectif était de créer un délit spécifique pour sanctionner la perturbation de l'exercice de certaines libertés fondamentales, avec des garde-fous : il faut prouver une action concertée et l'existence de menaces. En plus de cet article existent d'autres dispositions pénales permettant de condamner les auteurs de violences ou menaces de violences. En définitive, si nous nous indignons face à tout ce qui fait obstacle à l'exercice de libertés, une majorité du groupe RDSE considère qu'il n'est pas opportun d'élargir le champ d'application de l'article 431-1 du code pénal. de l'amendement Prince, qui ont obtenu l'avis favorable de la commission des lois ce matin, ne permettent pas de lever toutes nos inquiétudes. Leur adoption rajouterait en effet un risque d'instabilité jurisprudentielle, en insérant les notions d'« obstructions ou intrusions En outre, elles ne restreignent pas suffisamment l'application du délit d'entrave aux activités sportives ou de loisir. La notion d'activité « exercée dans un cadre légal » nous paraît trop vaste. Nous sommes toutefois désireux d'apporter une réponse utile au problème posé par ces « obstructions ou intrusions », qui sont une source d'angoisses pour nos concitoyens sur le terrain. C'est pourquoi nous proposons de différer ce débat, afin de nourrir une réflexion plus approfondie sur la façon de faciliter les modalités d'indemnisation des personnes lésées par ces comportements d'obstructions très pénalisants. Cela permettra d'ailleurs de mieux associer les représentants des activités concernées, ainsi que les acteurs chargés de l'application du texte. Des voies de recours sont déjà prévues en matière commerciale et pourraient par exemple être étendues aux chasseurs en en s'inspirant de la jurisprudence du 5 juillet 2018 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci reconnaît ainsi que « l'impossibilité psychologique de pratiquer une activité de loisirs constitue un préjudice d'agrément indemnisable Ces pistes, comme d'autres que nous pourrions explorer, nous paraissent plus adaptées aux attentes exprimées. La parole

Dois-je rappeler que nous sommes le seul pays en Europe à dispose d'une police spécialisée de l'environnement, avec des effectifs de plus de 2 000 professionnels qualifiés ? N'oublions jamais que, si nous avons cette police rurale unique, nous le devons aux fédérations de chasseurs et de pêcheurs qui avaient créé elles-mêmes, voilà plusieurs décennies, une garderie spécialisée pour lutter contre le braconnage et les dégradations de la nature. C'est ensuite l'État qui en a fait le corps de fonctionnaires que nous connaissons aujourd'hui et qui est placé sous la double tutelle des ministères de l'écologie et de l'agriculture.

Cette police des territoires, des espaces naturels, agricoles et forestiers et de l'eau est aussi une demande forte et insistante des gestionnaires que sont les agriculteurs, les forestiers, les élus locaux et, bien sûr, les chasseurs et les pêcheurs. Tous demandaient que la police rurale ne soit pas le parent pauvre des politiques publiques. Il y a longtemps que la faiblesse des effectifs départementaux de la police de l'environnement inquiétait ceux qui exercent tous les jours ce travail sur le terrain. Les chasseurs, les pêcheurs et les maires ruraux ont été les premiers à demander que la police rurale retrouve des effectifs, des moyens et des prérogatives pour agir contre toutes les formes de dégradation ou de braconnage qui menacent la biodiversité et la vie dans nos campagnes. Chacun sait que la gendarmerie nationale, qui a fait un travail remarquable et permanent dans nos territoires ruraux, ne peut plus tout faire, compte tenu de

Toutefois, malgré tous ces renforcements, cela ne suffit pas pour prendre en compte les nouvelles formes de violence qui commencent à se développer dans nos campagnes. Comme mes collègues, je crois indispensable de faire évoluer le droit, afin que l'on puisse donner une réponse à de nouveaux types d'entraves qui se multiplient contre des activités tout à fait légales. Depuis peu, les actions violentes commises par des groupuscules antispécistes, animalistes ou véganes se sont multipliées et deviennent insupportables pour tous ceux qui sont respectueux des lois de la République. Au nom de quelle idéologie sectaire certains peuvent-ils se permettre d'entraver des activités totalement légales, en vertu d'un ordre moral qui leur appartient ? Les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les éleveurs, les bouchers et les poissonniers, comme bien d'autres ruraux, sont des femmes et des hommes qui méritent le respect et qui doivent pouvoir exercer leur passion ou leur métier sans la moindre menace, dès lors qu'ils pratiquent ces activités dans le respect des lois de la République. Cette radicalisation de groupes extrémistes de la défense animalière doit être prise en compte à l'échelon de la sécurité intérieure, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays. Bien sûr, cela ne doit pas empêcher chacun de pouvoir se nourrir comme il l'entend et, au nom de la liberté d'expression, de tenter, s'il le souhaite, de convaincre le maximum de ces concitoyens de changer leurs habitudes alimentaires. Néanmoins, cela ne peut se passer que dans le respect d'autrui et non avec des méthodes d'obstruction, des menaces ou des actes de violence qui doivent conduire l'État à une vigilance accrue et à une sévérité à toute épreuve, vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire

cette expression chère à Jean-Noël Cardoux est sans doute la parfaite illustration de ce texte, qui ne donne pas une définition assez stricte au regard de l'exigence constitutionnelle de précision et de clarté de la loi pénale. volet des critiques de la commission des lois me semble plus discutable, car je ne crois pas que, en l'état du droit, les dispositions législatives existantes soient suffisantes pour réprimer efficacement la majorité des infractions visées.

Si nous ne le faisons pas, nous allons au-devant de réactions incontrôlées de la part de citoyens pratiquant des activités légales et qui, ne se sentant plus défendus, auront envie de se faire justice eux-mêmes, ce qui serait la pire des situations.

de nous celles et ceux qui vivent et travaillent dans nos campagnes et exercent un métier ou une passion respectable, qui donne du sens à leur vie quotidienne et qui est un véritable mode de vie. Mes chers collègues, à nous d'être à la hauteur et de produire un texte qui réponde à cette attente de bon sens et mette un terme à l'activité de ces groupuscules sectaires qui méprisent la démocratie, fût-elle participative. La parole

en croire l'argumentaire de la droite sénatoriale, ces éléments de contestation, aujourd'hui parfaitement légaux, devraient être réprimés sous prétexte que « contrevenir à la loi, ce n'est pas nécessairement faire ce qu'elle interdit ; c'est aussi empêcher ce qu'elle autorise ». En somme, ces moyens d'action seraient davantage « l'expression de convictions que de droits Ne nous leurrons pas : il est proposé ici de brider toutes les pratiques venant témoigner du moindre soupçon de défiance à l'égard de l'ordre établi. De l'ordre CRCE avait demandé par voie de communiqué de presse le retrait de ce texte de l'ordre du jour. Après la loi gouvernementale répressive venue encadrer le droit à manifester

Sur la forme, en nous soumettant cette proposition de loi, Les Républicains se prêtent à un exercice juridique particulièrement curieux. Tout d'abord, ce texte est anticonstitutionnel et sera sans aucun doute retoqué par le Conseil des sages s'il est adopté. Ensuite, il vient dénaturer l'article 431-1 du code pénal, qui sanctionne les entraves à la liberté d'expression. Ce dispositif va donc à contresens du droit positif. Mes chers collègues, la philosophie liberticide et antidémocratique de ce texte est profondément inquiétante. Nous ne pouvons tolérer les entraves aux mobilisations citoyennes, dont la tradition s'inscrit dans l'histoire de la France français ! Pensez aux suffragettes, par exemple. Comment oublier que nous devons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen aux révoltes du peuple français contre ses élites ? Comment oublier que les congés payés ont été obtenus par les piquets de grève de 1936 ? Cela n'a rien à voir ! Comment oublier le courage et la persévérance de ces milliers d'étudiants qui ont fait plier le gouvernement Villepin sur le CPE, le Des écologistes aux étudiants de Nuit debout, en passant par les « gilets jaunes », nombreux sont les exemples de revendications citoyennes ayant nourri la culture politique de notre pays. Protester, manifester, faire entendre sa voix et ses convictions est une coutume bien française à laquelle nous ne sommes pas près de renoncer. Vous cherchez aujourd'hui à rendre inconciliables certains droits : le droit de grève et le droit de travailler, le blocus devant un supermarché le droit de consommer, le droit de manifester des lycéens et leur droit d'étudier, le droit de défendre les animaux et le droit de pratiquer la chasse à courre. Par votre vision manichéenne du monde, vous scindez la Nation en deux, avec, d'un côté, ceux qui se complaisent dans l'ordre établi, et, de l'autre, ceux qui militent pacifiquement pour le changement. La plupart des mouvements citoyens ne sont pas mus par la haine, la violence et le rejet de l'autre. Beaucoup usent des moyens d'action collective pour exprimer leur envie d'entrer dans une ère nouvelle, plus sociale et égalitaire, plus respirable et durable. Les revendications écologistes et féministes sont ces dernières années intrinsèquement liées à la désobéissance civile : faucheurs d'OGM, les ZAD de Notre-Dame-des-Landes et de Bure, les animalistes, les décrocheurs du portrait du président Macron, les grévistes pour le climat, les militantes protestant contre les féminicides Ce que vous souhaitez, somme toute, c'est une uniformisation de la société. Vous désirez une France où chacun pense de la même manière et, de préférence, comme vous. Au risque de vous décevoir, tant qu'une opposition parlementaire comme la nôtre existera, tant qu'une jeunesse sera prête à se lever pour ses idées, tant qu'une gauche sociale et écologique s'exprimera dans ce pays, vous ne parviendrez

la proposition de loi qu'il nous est donné d'examiner aujourd'hui vise à apporter une réponse plus efficace à des agressions qui se multiplient. En effet, depuis quelques années, de nouvelles menaces liées à des groupes extrémistes de défense de la cause animale sont apparues, occasionnant des attaques contre des boucheries ou des étals, des intrusions dans des exploitations agricoles, allant jusqu'à l'incendie d'un abattoir. Voilà qui n'est pas très pacifique Ainsi, au cours de l'année 2018, la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs a recensé une cinquantaine d'agressions. De même, les entraves à la chasse se sont multipliées : des permanences de chasseurs ont été saccagées, des interventions en forêt ont parfois présenté un danger pour les cavaliers ... J'ai moi-même reçu des menaces de mort en inaugurant une maison de la chasse, anonymes bien sûr, car ces gens ne sont pas très courageux ! Ces actes commis par des individus qui cherchent à imposer leurs opinions par la violence ou par l'intimidation ne sont pas acceptables.

Si les citoyens ont le droit d'exprimer leurs convictions au sujet du bien-être animal ou de la consommation de viande, en revanche, au sein d'un État de droit, aucun individu ne saurait imposer ses opinions au moyen de la force. Comme l'a rappelé notre collègue François Bonhomme dans son rapport, « la République respecte la liberté et les choix de vie de chacun de ses citoyens Face à la radicalisation de certains groupuscules, une réaction s'impose afin de mettre un terme à ces actes. Oui, contre ceux qui attaquent les boucheries ou s'introduisent dans les élevages, une plus grande fermeté paraît nécessaire. Oui, la volonté d'imposer ses convictions ou d'empêcher certaines activités par la force ou la menace doit être sanctionnée. Car la violence et l'intimidation n'ont pas leur place sur le territoire de la République. Face à l'évolution inquiétante des actes de ces extrémistes animalistes, véganes ou antispécistes, les auteurs de la proposition de loi ont souhaité modifier l'article 431-1 du code pénal, afin d'apporter une réponse plus efficace et plus ferme à deux types d'infractions les violences, les menaces et les dégradations dirigées contre des boucheries ou des abattoirs au nom de la défense de la cause animale, d'autre part, les entraves à la chasse qui ont lieu régulièrement dans nos forêts domaniales. Toutefois, ce texte pose plusieurs problèmes. En premier lieu, la formulation du texte pourrait susciter des difficultés en raison de son caractère très général, au regard de l'exigence constitutionnelle à la fois de clarté et de précision de la loi pénale. En second lieu, des questions ont été soulevées sur l'utilité d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans la mesure où diverses incriminations pénales peuvent déjà être utilisées pour sanctionner ce type de comportements- peut-être ne sont-elles pas convoquées assez souvent. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires permettent de poursuivre les entraves, mais aussi les menaces, les violences et les dégradations. Toutefois, nous constatons que les amendements de précision qui ont été examinés en commission

nous risquons de voir se développer des actions d'autodéfense qui seraient préjudiciables à la vie démocratique. La parole

quels sont précisément les personnes et les actes visés par ce texte ? Après le débat approfondi que nous avons eu la semaine dernière en commission des lois, il me semble que nous avons une réponse

Je ne méconnais pas l'actualité de ces problématiques et, comme un certain nombre des orateurs qui m'ont précédé, je condamne avec la plus grande force tous ces délits ou contraventions au droit qui posent des difficultés très importantes dans le pays. Le débat en commission mercredi dernier a été nourri et, comme moi, plusieurs membres du groupe UC ont fait part de leurs réticences sur ce texte. Bien entendu, les critiques formulées ne visent en aucun cas à légitimer telle ou telle forme d'action militante, mais il nous paraît indispensable que, sous couvert d'intentions louables, nous ne portions pas atteinte aux libertés publiques de manière disproportionnée. Or la rédaction initiale du texte était extrêmement peu précise, visant à faire entrer dans la définition du délit d'entrave le fait d'empêcher « tout évènement ou toute activité autorisée par la loi ». Il convient de rappeler à ce stade que c'est de notre code pénal qu'il est question cet après-midi. Celui-ci, sans être sacré, présente un caractère particulier et la formulation très générale, pour ne pas dire vague, de l'infraction que je viens de rappeler risquait sans doute d'être jugée incompatible avec le principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines.

Cet après-midi, il ne s'agit pas de modifier le code de l'environnement, comme c'était le cas avec l'amendement créant un délit spécifique d'entrave à la chasse adoptée par le Sénat, au mois d'avril dernier, lors de l'examen du projet de loi Biodiversité. Que l'on soit pour ou contre cet amendement défendu par Jean-Noël Cardoux, il avait au moins le mérite de la clarté : il tendait à définir un délit qui ne concernait que l'entrave à la chasse, et il n'était pas question de modifier le droit pénal et le code pénal. L'ensemble de ces éléments m'a conduit, avec plusieurs de mes collègues, à voter contre cette proposition de loi en commission. L'opposition que nous avons formulée alors n'a pas été vaine, puisque, aujourd'hui, notre collègue Jean-Paul Prince, en collaboration avec l'auteur du texte, Jean-Noël Cardoux, et avec notre rapporteur, François Bonhomme nous propose une nouvelle rédaction de l'article unique de la proposition de loi. Celle-ci lève de nombreuses imprécisions ; elle permet également d'opérer une distinction salutaire entre les activités professionnelles, qu'elles soient commerciales ou artisanales, et les activités de loisir, comme la chasse. Il est normal que la peine encourue lorsqu'il s'agit d'entraver une activité de loisir soit plus faible que lorsqu'il s'agit d'empêcher d'exercer une activité professionnelle. Lors de la réunion du groupe Union Centriste aujourd'hui, nous avons largement débattu de ce texte et, à juste titre, de nombreux collègues ont fait valoir leur indignation face à des comportements violents à l'égard de certains commerçants ou à l'égard de chasseurs, comme face à l'intrusion dans des propriétés privées, comme des exploitations agricoles, ou à des actes de vandalisme. Tous ces actes sont insupportables, et nous les condamnons évidemment. Quelle que soit la cause que l'on défend, on ne peut

Il est donc important de faire la part des choses. Nul besoin de légiférer aujourd'hui pour pouvoir poursuivre un militant qui aurait eu un comportement violent envers un boucher ou qui aurait incendié un poulailler. Nul besoin non plus d'un nouveau texte pour condamner l'auteur d'actes de vandalisme dans une exploitation agricole ou de vols d'animaux, ou celui qui viendrait dégrader une permanence parlementaire. L'ensemble de ces comportements tombe déjà, et c'est heureux, sous le coup de la loi pénale.

cette proposition de loi, si l'amendement proposé par Jean-Paul Prince est adopté. Un certain nombre de nos collègues nous ont indiqué vouloir s'abstenir. À titre personnel, je voterai ce texte amendé. Avant de conclure, je tiens à attirer l'attention de la Haute Assemblée sur un point qui me semble extrêmement important.

Nous pouvons tous, cela a été dit, souscrire à cet objectif. En effet, il ne faut pas oublier que l'histoire nous a montré que c'est souvent par des violences interdisant aux citoyens l'exercice de leurs droits et de leurs libertés constitutionnelles que des groupes ou des partis extrémistes ont imposé leur domination à des sociétés jusque-là démocratiques. De fait, nous désapprouvons les manifestations qui font entrave à des activités légales et à l'expression de libertés publiques. Cela étant, la seule question que nous devons nous poser, en tant que législateur, est celle de savoir si les modifications proposées sont ou non pertinentes au regard du droit existant. Or, premier constat, l'ensemble des textes existants permet déjà de sanctionner les actes de violence. L'article 431-1 est sur ce point relativement clair. Deuxième constat, les modifications proposées aboutissent, à notre avis, à ne plus définir strictement le délit d'entrave, cela a été souligné à plusieurs reprises, ce qui est contraire au principe de l'intelligibilité de la loi. En effet,

À ce problème de preuve s'ajoute la complexification de la qualification. Le droit en vigueur vise le délit d'entrave,

Troisième constat, les modifications semblent contraires au principe de légalité criminelle, qui exige la définition par la loi des comportements répréhensibles. En envisageant de réprimer ce qui viendrait « empêcher », qui plus est « par tous moyens », « tout évènement ou toute activité » dont on suppute qu'ils seraient autorisés parce que non expressément interdits, les auteurs de la proposition de loi invitent le législateur à incriminer l'ensemble du champ social.

de l'imperfection des textes répressifs et de l'opportunité de sanctionner un comportement déviant inédit, ce principe constitue une garantie contre l'arbitraire. L'article 114-4 du code pénal

de l'actuel article 431-1 du code pénal semblent mesurés, l'extension du domaine, telle que la propose le texte, viendrait à dénaturer le sens originel et introduirait dans notre droit un délit d'entrave général disproportionné, voire dangereux, qui viserait toute contestation collective. Cette proposition de loi est une nouvelle illustration de ce que le doyen Carbonnier appelait « l'effet macédonien », c'est-à-dire une réaction générale et abstraite face à une agression concrète et particulière de moins grande ampleur. Cela appelle de notre part une grande vigilance, car cette proposition de loi témoigne de ce phénomène, par lequel le législateur est sollicité en vue de restreindre la liberté de tous. Cette vigilance s'est, je crois, largement exprimée lors de l'examen du texte en commission des lois, et c'est plutôt rassurant sur notre institution. Eu égard à ces éléments, et parce que nous désapprouvons, comme les auteurs de ce texte, les actes violents et répréhensibles qui ont eu lieu contre des activités légalement autorisées, il nous semble plus opportun il nous semble plus opportun et proportionné de reprendre la proposition faite par notre rapporteur en commission des lois : préciser que l'entrave réprimée à l'article 431-1 du code pénal prendre la forme de menaces, coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, mais aussi d'actes d'obstruction ou d'intrusion, ce qui permettra de qualifier un peu plus le terme « entrave ». C'est dans cet esprit que nous avons déposé l'amendement que nous examinerons tout à l'heure. En revanche, nous groupe sera opposé à toute extension du champ d'application de l'article 431-1 qui pourrait signifier une criminalisation de l'ensemble du champ social, car cela reviendrait à avaliser l'inversion du rapport entre le principe de légalité criminelle et le comportement

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, il y a plus d'un siècle, l'écrivain britannique Chesterton l'avait prophétisé : « Un temps viendra où l'on devra tirer l'épée pour défendre le droit de dire que, l'été,

La proposition de loi que nous examinons prévoit d'étendre le délit d'entrave, afin de pouvoir sanctionner toute action qui empêcherait l'exercice d'une liberté ou d'une activité autorisée par la loi.

On marche sur la tête ! Je remercie donc Jean-Noël Cardoux, auteur de la proposition de loi, qui, par ce texte, rappelle deux évidences qui sont au fondement de notre démocratie la liberté commence là où s'arrête celle des autres et que la France est un État de droit. Cela signifie que, dans notre pays, on ne doit pas pouvoir empêcher ce qui est autorisé. Deux actions légales sont visées de manière de plus en plus récurrente : l'élevage et les activités de boucherie, mais aussi, plus largement, toutes les activités liées au monde rural. Dans mon département, je suis régulièrement interpellé par des éleveurs ou des exploitants victimes d'intrusions dans leur exploitation agricole par des individus ou des associations anti-viande, notamment. Non seulement ces activistes sont pris en flagrant délit de violation de propriété et de non-respect des règles de biosécurité, mais ils font du mal à nos éleveurs et à notre agriculture. Or c'est grâce Or c'est grâce à nos éleveurs que la France est encore une puissance agricole de premier plan, représentant à elle seule 17 % de la production européenne. Je rappelle que, dans chaque filière agricole, il y a des hommes et des femmes qui font bien leur travail et qui ont à coeur de nourrir la population.

Sur le terrain, monsieur le secrétaire d'État, la situation est tendue. Certains agriculteurs, excédés, menacent d'intervenir eux-mêmes en séquestrant les individus. Imaginez les drames qui pourraient advenir ! Nous devons donc tout faire pour protéger

devons donc enrayer la montée en puissance de ces pratiques et poursuivre leurs auteurs avec fermeté. Le monde rural ne saurait être victime d'intimidations sans protection de notre part. Il nous faut agir. En tant que législateur, nous sommes les garants des droits et des libertés de valeur constitutionnelle. À ce titre, il apparaissait fondamental qu'une clarification juridique soit apportée, pour mieux définir le délit d'entrave et permettre des poursuites au civil et au pénal. La présente proposition de loi repose donc sur le constat que si les interdictions sont en règle générale assorties de sanctions, le législateur réprime plus rarement le fait de faire obstacle à ce que la loi autorise.

L'article unique du texte prévoit ainsi de modifier la définition du délit d'entrave. Mes chers collègues, le groupe Les Républicains votera majoritairement en faveur de ce texte. Je vous invite à faire de même. Là où la liberté dans notre pays est menacée, il est de notre responsabilité de la protéger. La discussion

La commission des lois a eu, au cours de deux séances successives, des débats approfondis sur ce texte. La semaine dernière, nous n'étions pas parvenus à un accord avec l'auteur de la proposition de loi, l'amendement qui avait été adopté en commission n'ayant pas paru suffisant à la majorité des membres

loi. Nous pensons que, si vous adoptez l'amendement que nous avons accepté en commission des lois ce matin et sur lequel notre rapporteur a

comme beaucoup d'entre nous, de souscrire à des dispositions qui les remettraient en cause. Madame Benbassa, faire valoir ses convictions ne permet pas tout. Quand vous faites obstacle à une activité autorisée par la loi, voire encadrée par elle, comme la chasse, vous ne faites pas usage de votre liberté d'expression,

Ces dernières années, les exploitations agricoles ont subi des intrusions illégales de plus en plus fréquentes. Force est de constater que seule la violation de domicile est invocable. Or celle-ci n'est pas suffisante. Ces intrusions peuvent avoir des conséquences parfaitement dommageables, qui vont bien au-delà d'une pénétration dans un domicile. Les agriculteurs se trouvent donc trop souvent démunis face à la réponse apportée à ces intrusions. Cet amendement tend à corriger cette situation en instaurant une infraction spécifique pour le monde agricole. Il s'agit de garantir le respect des bons usages en termes de biosécurité, de permettre la poursuite de toute personne

Ce que vivent les agriculteurs concernés est totalement inacceptable. Il est donc absolument nécessaire de renforcer les dispositions législatives applicables en la matière.

satisfait. Notre droit pénal permet déjà de sanctionner le fait de s'introduire et de se maintenir dans un local industriel, commercial ou professionnel sans l'accord de son propriétaire. C'est l'article 226-4 du code pénal. Le fait d'inciter autrui à commettre cette infraction peut également être sanctionné, sur sur le fondement de l'article 121-7 du même code. Les violences, les destructions et les dégradations qui seraient commises à l'occasion d'une intrusion dans des locaux professionnels peuvent aussi être poursuivies et sanctionnées. Il me semble donc que nous disposons déjà d'un arsenal législatif complet et suffisamment dissuasif pour lutter contre les intrusions dans les bâtiments agricoles. L'enjeu est d'appliquer avec détermination les dispositions en vigueur, monsieur le secrétaire d'État. La chancellerie a d'ailleurs donné au parquet des instructions de fermeté pour le traitement de ces affaires. J'ajoute que, de manière plus générale, il n'est sans doute pas de bonne pratique législative de multiplier dans le code pénal les incriminations spécifiques, comme c'est le cas en l'espèce.

viens de faire référence. L'instruction pénale de février 2019 qui a été donnée par la chancellerie aux parquets de France concerne les mouvements animalistes radicaux

parfois violents, dont sont victimes certains de nos compatriotes. Je pense notamment aux agriculteurs, aux bouchers, aux chasseurs et aux pêcheurs, mais d'autres sont également visés. Cet amendement tend à donner une définition plus précise et plus explicite de l'entrave. De plus, le régime de peines est modifié : les entraves aux activités professionnelles, commerciales, artisanales et agricoles sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, que les actes d'obstruction aux activités sportives et de loisirs sont punis de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende. En démocratie, chacun est libre de ses opinions,

C'est pourquoi j'espère que la présente proposition de loi sera votée par le Parlement et que ces comportements inacceptables disparaîtront, au profit du débat démocratique et du respect mutuel.

ou de la compléter. La rédaction de la proposition de loi telle qu'elle nous est présentée est trop imprécise, et son adoption serait de nature à remettre en cause la liberté d'expression, de réunion, de manifestation que l'article 431-1 du code pénal a justement pour objet de protéger.

en commission et en séance, en réduisant l'imprécision du texte, afin de ne pas porter atteinte au principe constitutionnel de précision et de clarté de la loi pénale, tout en restant fidèle aux objectifs. Je rappelle simplement qu'il comporte trois avancées. Tout d'abord, il vise à préciser les modalités de l'entrave qui peut être opérée en visant les actes d'obstruction ou d'intrusion. Cet ajout permettrait précisément de réprimer efficacement ces entraves constatées sur le terrain. Ensuite, il tend à mentionner les entraves aux activités commerciales, artisanales et agricoles. Il s'agit d'une formulation plus précise, qui fait référence à tous les évènements et à toutes les activités autorisés par la loi. Enfin, il a pour comme cela a été dit par le président de la commission, un délit d'entrave aux activités sportives et de loisirs exercées dans un cadre légal, mais avec un quantum de peines plus réduit. Il paraît en effet pertinent de sanctionner plus lourdement les entraves aux libertés fondamentales que sont les activités économiques que de punir les entraves à la chasse. Telles sont les raisons pour lesquelles j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 2 rectifié

d'obstruction et d'intrusion, les éléments constitutifs de l'infraction restent imprécis et paraissent donc contraires au principe de la légalité des délits et des peines. La jurisprudence indique d'ailleurs que le délit d'entrave est suffisamment défini par les termes de « violences » ou de « voies de fait De surcroît, la création d'un délit d'entrave pour certaines activités économiques, comme le vise l'amendement, n'est pas forcément cohérente, puisqu'il existe déjà un délit d'entrave à l'exercice de la liberté du travail. La disparition de toute référence à des actes précis pour caractériser l'entrave apparaîtrait donc également contraire à la Constitution.

On fragilise l'une des plus belles filières semencières européennes, la filière française, qui représente pratiquement 12 000 emplois et plus de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Monsieur le secrétaire d'État, je vous demande très sincèrement de revoir

Lorsque le juge décide que voler le portrait du Président de la République dans une commune, finalement, c'est défendre une cause juste, cela pose un problème ! C'est lamentable

De plus, mais c'est un débat récurrent que nous avons de part et d'autre de cet hémicycle et au-delà, croire que créer de nouvelles peines ou les augmenter suffira

l'heure lors de la discussion générale : « La proposition de loi déposée par le sénateur Jean-Noël Cardoux il y a quelques mois avait justement un objectif plus large et nous paraît être le bon cadre pour un examen par les assemblées de ces questions. En parallèle, il importera de caractériser finement

ainsi que des actes d'obstruction, sans plus de précisions, ayant pour effet d'empêcher le déroulement d'activités sportives ou de loisir.

près de 5 000 veaux. Or une partie de la ferme a été incendiée, avec des préjudices graves. Récemment, des engins qui travaillaient à la mise en place d'une serre à tomates complètement écologique,

dans notre démocratie, mais la République, c'est la liberté et non la violence. C'est non par des gestes

que la loi actuelle suffisait, mais cette proposition de loi, à mon sens, conforte la loi actuelle en apportant des réponses plus précises aux actes d'entrave.

Nous nous opposons bien évidemment à la logique d'une telle proposition, qui, loin d'atténuer les effets du texte d'origine, vise la même logique répressive et porte atteinte aux libertés fondamentales. Va-t-on vraiment punir les citoyens qui forment un blocus autour des supermarchés afin de dénoncer pacifiquement le consumérisme de nos sociétés ? Va-t-on emprisonner les militants de la cause LGBT qui mèneront des actions lors des matchs de foot, afin de faire cesser les chants homophobes dans les stades ? Ces actions ne constituent en rien un danger pour notre population et ne sauraient être réprimées de la sorte. Elles sont, au contraire, d'utilité publique et permettent d'informer et de conscientiser nos compatriotes.

le rapporteur soutient l'amendement présenté par M. Prince. L'amendement de mon groupe ne sera donc pas suivi, et la question sera celle du vote final. Monsieur le secrétaire d'État, pour une fois, je suis d'accord avec vous : ce texte est globalement inutile.

l'article 431-1 du code pénal que vous donnerez à la police les moyens d'enquête qui lui manquent. Car le vrai sujet, c'est bien celui-là. Par ailleurs, cette proposition de loi est dangereuse, car elle est attentatoire à nos libertés

dans une région où l'on pratique la chasse à courre, mais où les chasseurs font la différence avec la chasse à tir. Si nous appliquions ce nouvel article 431-1, le simple fait de se promener dans une forêt de l'ONF, par ailleurs louée